madame la ministre, mes chers collègues,

voter pour. Acte est donné de cette mise au point. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin concerné. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024 est parvenue à l’adoption d’un texte

Trésor (DGT) diminuent de six ETPT. Toutefois, nous nous félicitons de la préservation des emplois consacrés au réseau économique à l’étranger.

Après deux années de hausse des effectifs conformes à nos recommandations, l’année 2025 marque un retour en arrière, puisque trois ETPT seront supprimés, alors même que le champ d’action de la DGCCRF se diversifie. Les opérateurs de la mission prennent également largement leur part dans le redressement de nos finances publiques. Nous avons mis l’accent, dans nos travaux, sur le cas d’Atout France, dont la baisse importante des crédits et des emplois semble traduire l’amorce de la fusion avec Business France

Sont notamment concernés les secteurs de la sidérurgie, du papier ou encore de la chimie. Depuis plusieurs années, la hausse du prix du quota carbone conduit à une hausse mécanique du coût de la compensation. En 2025, elle atteint plus d’un milliard d’euros, soit une baisse de 23 millions d’euros par rapport à la loi de La deuxième évolution concerne Bpifrance. Nous nous félicitions, l’an dernier, de la création, dans le programme 134, d’une ligne budgétaire consacrée au financement des actions d’accompagnement des entreprises de Bpifrance. Or celle ci est purement et simplement supprimée dans le PLF pour 2025, ce qui constitue un retour en arrière du point de vue du contrôle du Parlement sur les financements de Bpifrance.

Madame la ministre, si nous souscrivons à l’objectif de décarbonation de notre économie que vise à atteindre cet amendement, nous déplorons la méthode retenue par le Gouvernement, qui nuit considérablement à la lisibilité de nos débats. Au regard de l’ampleur des montants annoncés, il eût été préférable que le Gouvernement fasse l’effort d’inscrire ces crédits dans le texte initial. Un sujet a particulièrement retenu notre attention lors de nos travaux. Je fais ici référence au désengagement de l’État du financement des pôles de compétitivité. En effet, l’enveloppe de 9 millions d’euros consacrée à ces pôles a elle aussi été supprimée dans le PLF. Les pôles de compétitivité ont pourtant fait la démonstration de leur intérêt pour le développement du tissu économique local et l’investissement privé dans la recherche et développement. Ce choix nous semble d’autant plus surprenant dans un contexte où le Gouvernement affirme vouloir engager notre pays dans la voie de la réindustrialisation. Nous vous présenterons tout à l’heure un amendement, partagé par l’ensemble des travées de cette assemblée, visant à rétablir cette ligne budgétaire. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en complément de l’intervention de mon collègue Thierry Cozic, j’aborderai pour ma part l’état du déploiement de la fibre optique, puis les compensations des missions de service public au groupe La Poste, avant de m’attarder sur la fusion d’Atout France et de Business France annoncée par le Gouvernement, sur laquelle nous sommes très réservés.

Ces RIP sont mis en œuvre dans le cadre de projets portés et financés par les collectivités territoriales. Les crédits du programme 343 subventionnant les RIP ont des effets positifs sur le déploiement dans les zones concernées. Toutefois,

À ce jour, seuls 87 % des locaux recensés en France sont éligibles à la fibre optique, c’est à dire raccordables. En outre, le taux de déploiement est très hétérogène sur le territoire. Surtout, les crédits consacrés au plan France Très Haut Débit ont déjà fait l’objet de coupes budgétaires massives en cours d’année 2024, et cette tendance devrait se poursuivre en 2025. Le PLF prévoit en effet une nouvelle diminution majeure des crédits consacrés aux RIP, en baisse de plus de 52 % par rapport à l’an dernier. Nous regrettons cette situation, qui risque d’affecter les collectivités locales. Celles ci devront, dans les cas où leur situation financière le permet, se substituer à l’État pour garantir le financement des projets. À défaut, cette situation se répercutera sur les opérateurs et leurs sous traitants, fragilisant ainsi le tissu La commission prend acte de cette baisse de crédits, justifiée par la situation dégradée de nos finances publiques. Toutefois, ce désengagement de l’État nous semble préoccupant et nuit à la crédibilité de la parole publique, puisque, rappelons le, le Gouvernement s’était engagé à déployer la fibre sur l’ensemble du territoire à l’horizon de 2025 ! Par ailleurs, nous vous présenterons tout à l’heure un amendement visant à sécuriser la concrétisation du plan France Très Haut Débit à Mayotte, qui, faute de crédits suffisants, n’est à ce jour pas garantie. Je poursuivrai en évoquant les compensations financées par la mission « Économie » et versées à La Poste au titre de ses différentes missions de service public. Je m’attarderai plus particulièrement sur le service universel postal et la mission d’aménagement du territoire de La Poste. La mission de service universel postal est compensée, en 2025, à hauteur de 500 millions d’euros, soit un montant stable par rapport à l’année dernière. Cela fait maintenant deux années que le PLF ne prévoit pas la part variable de 20 millions d’euros qui est censée être accordée en fonction du taux de lettres vertes effectivement livrées à J+3 par La Poste. Pourtant, les Pourtant, les résultats du groupe concernant ses délais de livraison sont conformes aux objectifs fixés. Nous vous présenterons donc un amendement visant à garantir que La Poste puisse bénéficier de cette part variable. Enfin, des questions majeures demeurent concernant la mission d’aménagement et de développement du territoire de La Poste en 2025. Cette mission essentielle consiste à maintenir des points de contact dans l’ensemble du pays. Elle fait l’objet d’un financement par le biais du Fonds postal national de péréquation territoriale.

Au total, 15 millions d’euros manqueront en 2025 pour atteindre le niveau de compensation cible de 174 millions d’euros. L’amendement que nous vous présenterons tout à l’heure tend à remédier à cette situation, et nous nous félicitons que le Gouvernement ait lui aussi pris cette initiative. Enfin, j’attire votre attention sur le projet de fusion entre Atout France et Business France, annoncé par le Premier ministre lors de son discours de politique générale en octobre dernier. L’ambition du Gouvernement est de réaliser des économies budgétaires, notamment par une mutualisation du réseau à l’international de ces deux opérateurs. Or les gains qu’est censée assurer cette fusion sont aujourd’hui très loin d’être démontrés. Cette réforme a été visiblement annoncée sans avoir été sérieusement préparée et sans que les acteurs concernés aient été consultés. Les missions d’Atout France et Business France ne se recoupent pas totalement. Atout France dispose d’une compétence métiers, illustrée par son action de développement de l’offre touristique sur le territoire français. Une fusion précipitée des deux opérateurs pourrait conduire à un affaiblissement de cette offre et avoir des conséquences négatives en termes de retombées économiques pour le secteur du tourisme. Par ailleurs, les suppressions d’effectifs au sein d’Atout France qui résulteraient d’une fusion pourraient impliquer des procédures de licenciement et reclassement coûteuses et sources de difficultés juridiques. Vous l’aurez compris, madame la ministre, nous sommes très sceptiques sur l’intérêt de cette réforme. La parole la commission des affaires économiques

de cette mesure, les crédits sont en réalité en baisse de 3 % en autorisations d’engagement et de 11 % en crédits de paiement. Pourtant, nous savons ici combien les missions de la DGCCRF sont plurielles. Ces dernières années, elles ont été considérablement étendues concernent aussi bien la régulation des influenceurs et le contrôle des négociations commerciales de la grande distribution que la lutte contre le. La DGCCRF s’est bien adaptée au développement de nouvelles pratiques de consommation. Il ne faudrait pas obérer ses efforts.

ou l’enrichissement des dispositifs de signalement SignalConso et RéponseConso. Concernant l’artisanat, la commission des affaires économiques se félicitait l’an dernier du lancement de la stratégie nationale pour les métiers d’art, à laquelle 3,4 millions d’euros de crédits étaient consacrés. Cette stratégie ne bénéficie d’aucun crédit dans le PLF pour 2025. En particulier, le label « Entreprises du patrimoine vivant » serait tout bonnement supprimé, alors qu’il est la vitrine de l’excellence et des savoir faire des artisans français à l’international. Les 1 500 entreprises labellisées sont connues du grand public et ont des savoir faire exceptionnels. Je pense aux verres Duralex, aux chaussures Repetto ou à la porcelaine Degrenne, pour n’en citer que quelques unes. Si nous en restions aux 200 000 euros de crédits actuellement consacrés à la gestion du label, aucune nouvelle entreprise ne serait susceptible de

de l’Union européenne. Toutefois, l’objectif de généralisation de la fibre optique jusqu’à l’abonné d’ici à la fin de l’année 2025 ne sera vraisemblablement pas atteint. En effet, le Plan

Dans la situation actuelle, si un effort généralisé est bien évidemment nécessaire, nous ne pouvons pas pour autant laisser subsister de fortes inégalités territoriales, à l’exemple, madame la ministre, de ce qui se passe dans le département de Mayotte, seul département français à ne pas disposer de la fibre optique.

est compromise par l’insuffisance de la compensation budgétaire versée au titre de la mission de contribution à l’aménagement du territoire. Alors que le contrat de présence postale territoriale, négocié avec les maires et les présidents d’intercommunalité, prévoit un financement de 174 millions d’euros par an, la compensation budgétaire prévue pour 2025 est de 105 millions d’euros.

d’environ 40 % par rapport à l’an dernier. Cette réduction concerne tous les secteurs, dans un contexte de réduction du déficit public. Alors que la Cour des comptes vient de dresser un bilan sévère des politiques publiques en faveur de l’industrie au cours de la dernière décennie, la commission des affaires économiques souhaite avant tout la pleine efficacité des dispositifs d’aide en vigueur.

Dans une logique de bonne allocation des deniers publics, je m’interroge aussi sur la suppression des dispositifs d’accompagnement non financier des entreprises par Bpifrance, alors que les études scientifiques montrent pourtant qu’ils ont un effet très positif, et plus important, à montant égal, que les aides financières

Enfin, le Gouvernement a déposé un amendement visant à abonder la nouvelle ligne dédiée à la décarbonation de l’industrie à hauteur de 1,5 milliard d’euros. Nous nous félicitons de cette réorientation, car il s’agit d’un enjeu majeur pour l’industrie de demain, et c’est bien en milliards d’euros que se chiffreront les besoins pour les prochaines années. Les 50 millions d’euros prévus dans le texte initial faisaient, à cet égard, bien pâle figure. Nous souhaiterions cependant des précisions sur les actions concernées et leur suivi, mais aussi sur les modalités de financement de cette enveloppe. Compte tenu de ces éléments, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable sur l’adoption des crédits de la mission « Économie ». Ce n’est pas, vous vous en doutez, la position du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, qui votera contre ces crédits.

pour avis. Madame la ministre, mes chers collègues, deux facettes de l’aménagement numérique de notre territoire ont particulièrement retenu l’attention de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Au premier semestre 2024, 89 % des locaux sont éligibles à la fibre optique, ce qui place la France, et nous pouvons nous en féliciter, dans le peloton de tête des pays européens.

Je déplore ce désengagement de l’État, qui oblige les collectivités territoriales à augmenter leur participation dans le déploiement des réseaux de fibre optique, alors qu’elles sont déjà fortement mises à contribution, à bien des égards, dans ce PLF.

au phénomène d’illectronisme dans les territoires, des conseillers numériques France Services ont été recrutés dans le cadre du plan France Relance. Malheureusement, malgré les engagements pris par l’État à son lancement, rencontre déjà des contrariétés budgétaires. En effet, les crédits alloués au déploiement des conseillers passent de 41 millions d’euros en 2024 à 27 millions d’euros en 2025. L’incompréhension face à cette baisse brutale des crédits est partagée par tous les acteurs du secteur Le désengagement de l’État pourrait conduire des espaces France Services à abandonner, faute de financement suffisant, la mise à disposition de conseillers numériques. Or ceux ci jouent un rôle pourtant essentiel auprès de nos concitoyens en situation d’illectronisme qui sont confrontés à la dématérialisation croissante des services publics.

les députés que la censure du Gouvernement serait une erreur historique pour notre pays. Les dirigeants d’entreprise, eux, l’ont bien compris. C’est la raison pour laquelle ils ont accepté, en grande partie, les efforts qui leur étaient demandés dans le projet de loi de finances pour 2025. Lucides sur les conséquences de la gestion calamiteuse des finances publiques et conscientes des risques d’une dégradation des conditions d’emprunt, les entreprises ont besoin de visibilité et donc, d’un nouveau budget pour l’année à venir. Il faut que nos collègues députés en soient conscients : la censure relèverait d’une irresponsabilité mortifère pour nos entreprises et pour notre pays. Une France sans budget, sans alternative et bientôt privée d’une partie de ses entreprises : sommes nous bien conscients de ce qui nous attend ? Les effets de l’incertitude politique et budgétaire se font déjà ressentir. Les taux d’emprunt de la France sur les marchés financiers ont plusieurs fois dépassé ceux de la Grèce. Le maintien de la notation de notre dette souveraine ne tient qu’au crédit accordé à l’actuel gouvernement pour réduire le déficit et redresser nos finances publiques. L’écart entre les taux d’emprunt français et allemand sur les marchés a atteint son plus haut niveau depuis 2012. La moitié des entreprises étrangères estime que l’attractivité du pays s’est dégradée. L’investissement est en panne. Les entreprises, prises dans l’étau du remboursement des prêts garantis par l’État (PGE) et de la hausse des coûts contraints comme l’énergie ou les assurances, licencient. On dénombre plus de 3 200 suppressions de postes par semaine, dont 1 219 dans les seules entreprises de moins de dix salariés. Ceux qui envisagent de censurer le Gouvernement doivent bien mesurer le poids de leur responsabilité, car ils semblent avoir oublié que la paralysie financière de la France retombera sur les entreprises, qui sont les seules à créer de la valeur. Or c’est cette création de valeur qui permet de financer nos services publics et nos politiques publiques, et de débattre de la répartition des crédits au sein des différentes missions de la deuxième partie de ce projet de loi de finances. Sans les entreprises, pas de salariés, donc pas de salaires nourrissant l’impôt sur le revenu et les cotisations patronales. Sans les entreprises, pas de bénéfices, donc pas d’impôts sur les sociétés. Sans les entreprises, pas de création de richesses en France, donc pas d’exportations pour combler le déficit abyssal de notre balance commerciale. Sans les entreprises, nous n’aurons même plus les moyens de réaliser des arbitrages budgétaires ; nous n’aurons plus que le souvenir douloureux d’avoir eu un jour le choix de définir nos priorités de dépenses et d’avoir gâché notre chance de nous en sortir. Initialement, j’avais prévu d’évoquer devant vous le financement des pôles de compétitivité et de soutenir notre commission des finances. Initialement, je comptais vous parler également de la suppression dans le programme 134 d’une ligne budgétaire dotée de 100 millions d’euros dédiés au financement des actions d’accompagnement des entreprises de Bpifrance. Je souhaitais rappeler l’importance de ce métier d’accompagnement, devenu une activité très importante de Bpifrance, qui permet d’accélérer la transition énergétique et environnementale et la digitalisation des petites et moyennes entreprises Or, aujourd’hui, du fait de l’éventuelle censure du Gouvernement, sans alternative pour le budget, l’enjeu ne sera même plus la croissance des PME. L’enjeu sera celui de leur survie. (CPME) l’a d’ailleurs clairement dit : « L’adoption d’une motion de censure signifierait l’ouverture d’une nouvelle période d’instabilité et un nouvel arrêt de l’économie qui tourne déjà au ralenti. […] La France et les Français, les entrepreneurs et les salariés, en paieraient lourdement le prix. Et nos entreprises seraient les premières victimes. » Si la censure est votée, nous allons en effet nous priver de toute création de richesses à cause d’une conjuration des irresponsables. La paralysie qui s’annonce est le produit d’une coalition des contraires. À la surenchère fiscale dont les entreprises ont été la cible principale s’ajoute une irresponsabilité des forces politiques. Les seuls bénéficiaires seront les extrêmes. Les seuls vaincus seront nos compatriotes les plus précaires, qui ne pourront pas se protéger de la faillite publique. Citoyens et entreprises sont pris au piège des jeux politiciens du PS, du RN et de LFI. Quel que soit le scénario envisagé ensuite, qu’il s’agisse de l’adoption du budget par ordonnance par le gouvernement démissionnaire ou de la reconduction du budget de 2024 par le truchement d’une loi spéciale, il nous sera impossible de redresser les finances publiques et de retrouver la confiance des marchés. Les investisseurs imposeront une prime de risque bien plus élevée. Le poids de la dette va asphyxier notre économie et, par conséquent, anéantir les marges de manœuvre dont nous disposions et dont nous avons débattu ensemble ici même. Alors que notre pays a besoin de mesures fortes lui permettant de ne pas reculer, nous ne pouvons pas nous offrir le luxe d’une crise financière se surajoutant à la crise politique et d’une défiance généralisée de la part des marchés qui financent notre dette. Les entreprises qui créent la richesse indispensable à la prospérité de tous méritent mieux. Les Françaises et les Français méritent mieux. La France mérite mieux. La

la mission « Économie » comprend une grande variété de programmes : « Développement des entreprises et régulations », « Statistiques et études économiques », « Plan France Très haut débit », « Statistiques et études économiques Stratégies économiques », ainsi que le financement des opérations patrimoniales le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Pour 2025, les crédits de l’enveloppe alloués à la mission « Économie » s’élèvent à 3,65 milliards d’euros en autorisations d’engagement et à 3,88 milliards d’euros en crédits de paiement, soit une baisse de 13,77 % en autorisations d’engagement et de 9,51 % en crédits de paiement, comme cela a déjà été rappelé. Malgré cette baisse, plusieurs mesures sont à la hauteur des politiques publiques visant à soutenir nos entreprises, mais aussi l’activité dans tous les territoires. Je pense ainsi au maintien de la compensation carbone pour prévenir le risque de délocalisation des industries. Le montant de la compensation carbone versée aux industries électro intensives des secteurs soumis à une forte concurrence internationale représentera ainsi en 2025 un budget initial de plus d’un milliard d’euros, et ce pour la deuxième année consécutive. Par ailleurs, afin d’accélérer le verdissement du tissu industriel français, deux leviers primordiaux sont mobilisés au sein de ce PLF. D’une part, le crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte continuera à soutenir l’implantation de chaînes de production impliquées dans les secteurs clés de la transition écologique : batterie, éolien, panneau solaire, pompe à chaleur. D’autre part, un dispositif de subvention des projets de décarbonation dans l’industrie destiné aux cinquante sites industriels les plus émetteurs sera lancé en 2025. Ainsi, pour la première fois, la programmation pour 2025 comportera une ligne de financement pour la décarbonation de l’industrie de 50 millions d’euros. La DGCCRF continuera également, en 2025, d’être mobilisée sur les problématiques de relations commerciales. Cela se traduira notamment par le renforcement des contrôles des pratiques commerciales des influenceurs, des sites de livraison directe, de modes éphémères ou de produits présentant un danger, ce dont nous pouvons nous féliciter. Toutefois,

La généralisation de la fibre optique est indispensable à la résorption des fractures numériques. La fibre constitue d’ailleurs souvent un élément d’attractivité pour les territoires. Nous Nous proposerons donc et soutiendrons les amendements visant à rehausser les moyens alloués à ces actions, en particulier ceux qui sont fléchés pour Mayotte. Ensuite, la baisse des crédits alloués aux dispositifs des conseillers numériques France Services est inquiétante. Elle fera passer le nombre de conseillers numériques de 4 000 à 1 500 en moyenne, alors que le dispositif a déjà permis plus de 4 millions d’accompagnements. Le groupe RDPI proposera ainsi de rehausser les moyens dévolus à ces conseillers. En conclusion, malgré certaines baisses de crédits de la mission « Économie plusieurs mesures sont à la hauteur des objectifs défendus et s’articulent avec l’ensemble des politiques publiques visant à soutenir nos entreprises, mais aussi l’activité dans tous les territoires. Le groupe RDPI votera donc ces crédits.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, Michelin, ArcelorMittal, Valeo… Si ces plans sociaux ont des résonances nationales, d’autres, moins médiatisés, fragilisent le tissu économique de nos territoires. cas en Loire Atlantique, avec les fermetures de Systovi, ou les restructurations de Saulnier Duval, General Electric, Goodyear, Cargill et, je le crains, bien d’autres. Entre 100 000 et 200 000 emplois sont ou seront détruits dans les prochaines semaines. C’est dans ce contexte aggravé par une crise politique majeure

au vu des actualités économiques. Ce n’est pas en s’attaquant à nos capacités à produire de la richesse que nous contribuerons à redresser nos finances publiques. Bien au contraire.

trouvent leur pertinence. Le désengagement de l’État du financement des pôles de compétitivité, pourtant moteurs de croissance, fragilise les tissus économiques locaux au moment où nos collectivités locales vont perdre leur capacité à investir. Sur l’industrie, pendant que les ministres successifs se gargarisent de « souveraineté industrielle » et de « réindustrialisation », les crédits sont en baisse de 39 % hors compensation carbone. Ce choix suscite des interrogations sur la cohérence politique entre ce qui est exprimé par votre gouvernement et la réalité brute. matière d’inclusion numérique, la baisse de 33 % des crédits pour l’accompagnement des personnes isolées par France Services fait supporter ce coup de rabot budgétaire aux publics les plus fragiles. Nous défendrons des amendements tendant à maintenir des moyens nécessaires à la poursuite de cette ambition d’égalité. Nous regrettons l’absence de révision du Fonds territorial d’accessibilité. Vous proposez la suppression d’une mesure facilitatrice sans proposer de solution de remplacement pour permettre l’accès de tous aux établissements recevant du public, en premier lieu nos petits commerces de proximité. l’économie sociale et solidaire est, en l’état, sous dotée. Nous soutiendrons l’amendement de notre collègue Michel Masset visant à consolider un secteur économique durable. Madame la ministre, nous déplorons le manque de moyens alloués à cette mission au regard des importantes difficultés des entreprises dans cette période troublée. le président de la chambre de commerce et d’industrie de mon département m’appelait, inquiet de la situation politique de notre pays. Il me prédisait les pires catastrophes alors même que notre territoire compte parmi les plus dynamiques de France. Les vœux de réindustrialisation et de consolidation de notre économie ne se concrétiseront qu’avec un accompagnement public à hauteur des enjeux. C’est aussi par l’investissement et un soutien massif à la recherche, à nos entreprises et à nos collectivités locales que l’État pourra, grâce à des dynamiques économiques renouvelées, s’assurer de nouvelles rentrées fiscales. Vous l’aurez compris, le budget proposé ne nous satisfait pas. Pourtant, fidèle à ces principes, le RDSE réserve son vote en privilégiant un débat constructif, dans l’intérêt de nos concitoyens. Je crains – hélas ! – que ce ne soit pas le principal souci de nos collègues députés à la veille de la chute annoncée du Gouvernement. À titre personnel, bien que ne partageant pas les orientations poursuivies depuis sept années par les gouvernements qui se suivent et se ressemblent, je regrette profondément ce pas vers le désordre et l’inconnu. Ce n’est pas digne de partis politiques qui aspirent au gouvernement de la France !

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en cette séquence politique inédite, gardons, s’il vous plaît, à l’esprit que c’est avec le monde économique que nous parviendrons à redresser un budget, et non sans lui. Compétitivité des entreprises, stratégie économique, industrialisation : cette mission « Économie » est au cœur de la réflexion sur la trajectoire que nous souhaitons pour la France. Elle soulève une question clé : politique d’austérité ou soutien ciblé au monde économique pour éviter une récession ? de budget, construit en un temps record, traduit une position hésitante de Bercy, sans réelle vision de long terme, attendue pourtant par les acteurs économiques. Si nous comprenons les contraintes actuelles, nous regrettons l’absence de réelles dispositions contracycliques qui permettraient d’affirmer un soutien renforcé à l’industrie et, plus largement, notre confiance envers le monde économique, levier essentiel pour accompagner la nécessaire rigueur budgétaire. Nous saluons toutefois plusieurs mesures positives, comme la rationalisation des crédits de dispositifs jugés inefficaces, le maintien des garanties de Bpifrance, le soutien à Business France pour accompagner les exportations ou les politiques de protection du consommateur. La semaine dernière, à Limoges, le Premier ministre rappelait avec justesse qu’un grand pays, c’est un pays qui reste une terre de production. Cette ambition essentielle pour l’industrie et l’innovation ne trouve pas un écho suffisant dans ces orientations budgétaires, ce qui appelle un certain nombre d’observations. Alors qu’une dynamique de réindustrialisation commençait à produire ses effets grâce à une hausse significative des crédits depuis 2023, nous observons avec préoccupation une baisse de près de 20 % des crédits du programme 134, dont une réduction de 11 % pour l’action n° 23 « Industrie et services », et, plus exactement, de 39 % si l’on si l’on exclut la compensation carbone. Par ailleurs, nous regrettons le manque de lisibilité de la politique industrielle, fragmentée entre le plan France 2030, le programme Territoires d’industrie et la mission « Économie ce manque de coordination compromet son efficacité et complique son pilotage. Autre point d’alerte, le message envoyé aux PME, qui apparaissent fragilisées par la suppression des lignes budgétaires dédiées à leur accompagnement et à leur restructuration, dispositifs pourtant efficaces et peu coûteux. enfin les coupes franches sur les pôles de compétitivité, qui favorisent l’innovation et profitent aux PME. Ces investissements stratégiques à long terme, peu coûteux, permettaient de développer des écosystèmes économiques vertueux, un réel soutien pragmatique aux côtés des collectivités locales.

Nous appelons de nos vœux un nouvel élan pour notre politique industrielle, au service de notre souveraineté économique et de notre attractivité.

pour plus de justice sociale, fiscale et environnementale, vous avez décidé de vous essuyer les pieds une nouvelle fois sur le Parlement en exigeant une deuxième délibération. Et

3 milliards d’euros supplémentaires sur les facteurs de gaz. Les gens ne trouvent pas d’emploi ? Nous en sommes à 300 000 emplois menacés ? Vous continuez à donner des cadeaux fiscaux, 200 milliards d’euros par an, sans vouloir une seule fois conditionner ces aides publiques et cet argent public ? Votre projet de budget pour

la mission « Économie » est le socle du développement industriel, de l’innovation et de l’entrepreneuriat de notre pays : un socle, c’est à dire une base, solide et stable, sur laquelle repose une structure, en l’occurrence la dynamique d’emplois de notre pays.

L’affaire Nestlé Waters a mis en lumière l’importance indiscutable de ses missions. Nous demandons une augmentation de cinquante équivalents temps plein pour que la DGCCRF puisse faire son travail et protéger les consommateurs. viens à l’économie sociale et solidaire. Comment avez vous osé couper un budget d’à peine 20 millions d’euros, qui concerne 15 % de l’emploi privé en France, 2,4 millions de personnes ? Je voterai donc l’amendement tendant à augmenter ce budget. Par ailleurs, avec plusieurs collègues de différents groupes politiques, nous défendons la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par leurs salariés. Pourquoi ? Parce que cela marche. Prenons l’exemple de Duralex, entreprise emblématique qui a connu quatre redressements judiciaires. Lors du dernier, les salariés n’ont pas cédé et, avec l’appui des élus locaux de tous bords, ils ont repris Duralex sous forme de société coopérative participative (Scop). Cela a permis de sauver les emplois, de préserver le savoir faire et de garantir l’avenir de l’usine. Ce projet a nécessité 10 millions d’euros. Heureusement que la région et la métropole ont pris cela en charge, parce que Bpifrance n’a pas privilégié la structure coopérative ! Ce fonds permettra peut être de sauver deux ou trois entreprises. Mais quand bien même il ne permettrait de n’en sauver qu’une seule, ce serait déjà une grande réussite. Je compte donc sur vous pour voter l’amendement concerné. Réduire les budgets de la mission « Économie », c’est fragiliser les fondements mêmes de notre dynamique économique collective. Faire et défaire, c’est toujours travailler, dit l’adage. Mais l’heure est grave. Ce que vous êtes en train de défaire va engendrer une crise sociale sans précédent. Et ce que vous êtes en train de faire est irresponsable compte tenu des enjeux climatiques planétaires.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission « Économie » subissent une baisse drastique de près de 14 % par rapport à 2024. Et, au sein de cette mission, le programme consacré à l’industrie enregistre une diminution de 12 %, alors même que le Gouvernement nous parle sans cesse de « réindustrialisation » comme priorité nationale. Comment expliquer une telle contradiction ? Ce programme est censé renforcer la compétitivité de notre industrie, accompagner les mutations économiques de nos entreprises et soutenir les territoires. Alors, pourquoi réduire précisément les moyens alloués à ces objectifs stratégiques ? Je note également la suppression pure et simple de la ligne budgétaire consacrée à la gouvernance des pôles de compétitivité, pourtant dotée de 9 millions d’euros en 2024. À l’heure où la désindustrialisation s’accélère, où la concurrence mondiale s’accroît et où les besoins en innovation territoriale s’intensifient, ce choix est purement incompréhensible. Dès lors, plusieurs questions se posent. Comment prétendre s’engager dans la réindustrialisation avec des budgets en baisse ? Comment prétendre soutenir nos industries alors que les plans sociaux se multiplient, touchant Michelin, Rougié dans notre département, Auchan, Valeo et tant d’autres ? Comment parler de reconquête industrielle

Enfin, la décarbonation de nos industries est essentielle, mais l’effort reste insuffisant et centré sur les grandes industries électro intensives. N’oublions pas nos TPE PME, qui sont le cœur battant de notre économie et de nos territoires. Elles aussi ont besoin du soutien face à la crise énergétique et à la compétition internationale. L’effort demandé est immense, mais les moyens alloués sont dérisoires. J’ai cherché, et j’avoue que je cherche encore, des motifs de satisfaction dans ce projet

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’étude de cette mission nous conduit à faire un constat simple, mais terrible la France est en récession ; nous sommes devant l’échec total d’une politique économique déjà bien entamée par le socialisme depuis 2012. Toutes les composantes de la croissance sont inférieures aux prévisions macroéconomiques du Gouvernement. On nous promettait en 2017 un « monde nouveau », le retour du sérieux et un langage de vérité devant les Français. Nous n’avons eu que le précipité du pire de l’ancien, mâtiné d’un mépris conformiste devant nos propositions raisonnables. Mais revenons au présent. Devant la dérive des comptes et de l’économie, le gouvernement précédent se défend péniblement, expliquant que le dérapage ne serait dû qu’à une mauvaise élasticité des recettes fiscales à la croissance. mois de décembre 2023, le gouvernement d’alors était au courant de l’affaiblissement inquiétant de l’économie. Bruno Le Maire, Élisabeth Borne, puis Gabriel Attal ont menti devant la représentation nationale et devant les Français. Après les déculottées électorales successives, nous sommes maintenant à l’heure des comptes et des efforts délirants demandés aux Français et aux entreprises. Depuis, la crise s’est aggravée : les entreprises n’investissent plus, les ménages consomment moins, les plans sociaux s’égrènent, charriant avec eux leur lot de drames sociaux et de dépenses publiques nouvelles. Le journal dresse la liste tragique des centaines d’entreprises qui déposeront le bilan en 2025. Ainsi, 160 000 emplois, et presque autant de familles, et bien plus d’emplois liés, vont bientôt disparaître. Toute la politique menée depuis sept ans n’a consisté qu’en paroles et en projets inaboutis. Même la Cour des comptes, que l’on ne peut pas accuser d’être un organe à la main du Front national, indique dans un rapport limpide que la politique de réindustrialisation n’a pas permis de progrès substantiels. L’emploi industriel baisse encore dans notre pays à des niveaux alarmants livré à une concurrence déloyale, à laquelle vous refuserez évidemment de vous attaquer. Encore une fois, nous proposerons au cours de la discussion des sources d’économies réelles dans le maquis des opérateurs d’État, dont les ressources ont considérablement augmenté depuis 2017. Loin d’apporter une technicité et une régulation efficaces, les agences et autorités publiques sont des trous noirs comptables et gestionnaires, où se perdent 80 milliards d’euros.

au retour à l’équilibre de nos comptes publics. Plus que jamais, pour sauver l’économie française et nos emplois, il faut une rupture : la rupture avec un système qui n’a jamais autant montré les preuves de sa faillite. Nos propositions sont sur la table. Il y a de grandes chances que vous les refusiez. Nous en prendrons acte. La parole

cette mission la mission du quotidien. Derrière ces grands mots, il y a en effet une réalité : des femmes, des hommes, de la passion, du labeur, du savoir faire, du travail, de la vitalité et de l’espoir quand cela va ; du chômage, de la pauvreté, de l’isolement, des vies malmenées – parfois brisées –, des petits patrons et des agriculteurs étouffés quand cela va mal. J’en passe, mes chers collègues.

La noblesse de cette mission, c’est de faire le pont entre le quotidien des gens et la souveraineté industrielle et numérique de notre pays. Je ne rappellerai pas le contexte financier et les conditions dans lesquelles ce budget a été rédigé ni les risques qui pèsent déjà sur la confiance dans notre économie. La situation que nous traversons est très grave et très incertaine. Le Gouvernement a élaboré un budget d’urgence. Il a décidé de faire porter l’effort pour un tiers sur une augmentation de fiscalité ciblée et pour deux tiers sur une baisse des dépenses publiques. La France étant l’un des pays les plus fiscalisés du monde – il faut en avoir conscience –, nous ne pouvons plus abuser du levier fiscal. Le « trop d’impôt » tue nos entreprises.

Quand on n’a pas d’argent, on ne dépense pas ! Arrêtons de vivre à crédit ! Cela vaut donc en particulier pour la mission « Économie », dont le groupe Les Indépendants propose une diminution de 2 % des crédits. C’est peu, mais nécessaire. Il ne s’agit pas de sacrifier tel ou tel service public

Je souhaite appeler votre attention sur trois sujets, en premier lieu sur l’industrie. Alors que les gouvernements successifs ne cessent de rappeler l’importance de réindustrialiser notre pays, la quasi totalité des lignes fléchées vers le soutien à l’industrie sont en baisse. Élu des Hauts de France, première région automobile française en termes de production de véhicules, je ne peux que relayer les inquiétudes des industriels et surtout des 56 000 salariés de la filière. Je prendrai moi aussi l’exemple des pôles de compétitivité. Comme la commission le préconise, j’invite le Gouvernement à les financer. Dans ma région, le pôle de compétitivité I Trans, pôle de compétitivité des transports, de la mobilité et de la logistique, est un atout considérable pour nos entreprises.

Toujours dans mon territoire, nous nous sommes battus pour sauver l’aciérie Ascoval, qui est devenue l’une des aciéries les plus modernes d’Europe. L’acier vert est vertueux. Mes chers collègues, madame la ministre, nous soutiendrons bien sûr l’amendement n° II 891, qui tend à créer une enveloppe complémentaire afin d’accompagner cette décarbonation.

Je tiens à saluer aussi tout particulièrement la mise à disposition d’une enveloppe de 16 millions d’euros pour le financement des raccordements complexes dans le domaine privé. C’est un réel besoin dans nos territoires, notamment dans nos communes rurales. de l’inclusion numérique, le désengagement est manifeste. Là encore, j’appelle le Gouvernement à réunir rapidement tous les acteurs du secteur, et ils sont nombreux. Nous devons rationaliser. Enfin, le troisième et dernier sujet est celui des compensations budgétaires versées à La Poste pour l’exercice de ses missions de service public.

fragiles. L’économie sociale et solidaire préserve le lien social et la vitalité de nos territoires. Ainsi, en Ariège, elle représente 12 % de l’emploi salarié et 4 200 emplois. Dans les zones rurales où le retrait des services publics et la désertification fragilisent l’économie locale, l’ESS reste le dernier rempart, assurant la protection des plus vulnérables. Les crédits de l’ESS avaient déjà été rabotés par l’annulation de 1,7 million d’euros en autorisations d’engagement et de 3,2 millions d’euros en crédits de paiement en 2024, et ce afin d’atteindre un déficit public

aurait pesé lourdement sur les communes rurales ou, pire, entraîné des fermetures de points de contact. La stabilisation de la subvention au titre de l’aménagement et du développement du territoire ne permet pas, cependant, de remédier à la sous compensation chronique de cette mission de service

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, madame, monsieur les rapporteurs spéciaux, mesdames, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à remercier les rapporteurs et les orateurs de groupe, ainsi que les sénatrices et sénateurs engagés sur cette mission, de leur travail d’analyse et de l’examen attentif des crédits de la mission. fil conducteur de mon intervention la façon dont le Gouvernement adapte son action pour financer ses priorités dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Les crédits de la mission « Économie » dans le projet de loi de finances pour 2025 s’élèvent à plus de 3,8 milliards d’euros en crédits de paiement, soit une diminution de 3 %, qu’il faut mettre en perspective avec l’évolution des crédits de la mission depuis la crise sanitaire. Le programme 134 « Développement des entreprises et régulations » a particulièrement porté les dispositifs d’urgence, les crédits concernés étant passés de 850 millions d’euros en 2021 à 6 milliards d’euros en 2023. Nous ne nous inscrivons donc pas dans une logique de rabot aveugle, ainsi que j’ai pu l’entendre tout à l’heure. Le PLF pour 2025 acte un retour à une situation normalisée, ce projet de budget contribuant au développement d’une stratégie soutenant la croissance durable et équilibrée de l’économie française. Premièrement, le soutien des acteurs économiques reste la priorité du Gouvernement, au service de la compétitivité, de l’accessibilité et de la durabilité de notre économie. Les aides aux entreprises en matière énergétique sont renforcées au profit de dispositifs visant à préparer notre économie à la transition écologique. Nous poursuivons notre politique d’accompagnement des entreprises électro intensives au travers du dispositif de compensation carbone. Celui ci est indispensable au maintien de leur compétitivité et à la prévention des délocalisations, et vient compenser les coûts liés au système européen des quotas d’émissions. Depuis plusieurs années, la hausse du prix du carbone conduit à une augmentation mécanique du coût de la compensation. En 2025, celle ci atteindra plus de 1 milliard d’euros, au profit notamment de la sidérurgie ou de la chimie.

Enfin, l’accès au guichet d’aide au paiement des factures d’énergie est élargi aux ETI. Ce dispositif, dont les conditions sont définies par un décret publié en 2024, vise notamment à compenser une partie des surcoûts d’électricité. une partie des surcoûts d’électricité. Le soutien que nous apportons à l’économie passe aussi par un effort accru pour renforcer l’accessibilité aux services publics. Nous affirmons le principe d’un soutien de l’État à La Poste

nous affirmons l’importance des 17 000 points de contact dans l’aménagement de notre territoire. L’accès aux réseaux de fibre optique répond également à cet enjeu d’aménagement, en permettant à nos concitoyens, aux entreprises et aux collectivités qui s’y raccordent de bénéficier de la qualité de service du très haut débit. Je suis sensible aux recommandations formulées par Frédérique Espagnac et Anne Catherine Loisier sur ce sujet. L’action de l’État s’inscrit déjà dans la continuité de plusieurs d’entre elles, comme le fait de sanctionner davantage les opérateurs lorsque ceux ci ne respectent pas les engagements qui leur sont opposables. Le budget proposé par le Gouvernement s’inscrit dans la continuité de l’année 2024 : il accompagne l’avancée des travaux de déploiement des réseaux d’initiative publique par les collectivités, et étend la politique de généralisation de la fibre optique, particulièrement dans les territoires les plus isolés.

En parallèle, nous poursuivons notre objectif d’amélioration de la compétitivité des entreprises par des soutiens qui se veulent ciblés. L’enjeu de souveraineté industrielle et numérique qui est placé au cœur de notre mandat requiert des entreprises compétitives et durables. En matière d’accompagnement à l’export des entreprises françaises et de développement des investissements étrangers, l’action déployée par l’État au travers de son opérateur Business France, en lien avec les régions, se poursuit au travers de la et de la. Par ailleurs,

Concernant les enjeux de l’économie du tourisme, à laquelle je suis particulièrement attachée, je suis consciente des inquiétudes que suscite le rapprochement entre Atout France et Business France. Je voudrais en quelques mots vous faire part de ma vision sur ce sujet.

Si les contours exacts de la réforme restent à préciser, le précédent Gouvernement avait fixé un certain nombre de principes, parmi lesquels la révision des missions et le renforcement des synergies avec d’autres opérateurs. ministre a pris, dans sa déclaration de politique générale, ce sujet comme exemple de la nécessité de regrouper les opérateurs de l’État exerçant des missions relativement proches, dans un objectif très clair de renforcement de l’efficacité de l’action publique. Pas sûr ! À la suite de cette déclaration et de ma prise de fonction, j’ai interrogé tous les acteurs du tourisme – collectivités territoriales, socioprofessionnels – pour connaître leurs attentes à l’égard d’Atout France, ainsi que leur perception de cette réforme. Tous s’accordent à dire qu’il y a matière à tirer parti de l’existence des réseaux des deux opérateurs à l’étranger pour porter de manière plus efficace l’action publique en matière de promotion de la destination France. Ils estiment Ils estiment qu’il est nécessaire de repenser globalement le maillage de ce réseau international, afin de l’orienter davantage vers les marchés à fort potentiel pour la France. Pour ce qui concerne les autres missions, les avis sont partagés sur la manière dont elles doivent être exercées. Tous reconnaissent néanmoins l’importance des missions conduites par Atout France, qu’il s’agisse de l’ingénierie, de l’observation ou des missions réglementaires. J’ai bien sûr également rencontré les agents d’Atout France et leurs représentants du personnel qui, dans cette période d’incertitudes, expriment des inquiétudes bien légitimes. Je tiens ici devant vous à saluer leur engagement et leur travail, qui a permis d’atteindre les objectifs qui leur avaient été fixés – 100 millions de touristes accueillis en France – et qui contribue ainsi à la relance de l’économie du tourisme, après l’une des plus graves crises que nous ayons connues. Dans ce contexte, j’ai souhaité lancer une mission de préfiguration,

ce qui fonctionne. Absolument ! Dans cette perspective, je serai particulièrement attentive à la préservation de l’expertise métier qui est aujourd’hui déployée par les agents d’Atout France. Au delà du lancement de cette mission de préfiguration, l’opérateur contribuera, comme les autres opérateurs de l’État, au redressement des finances publiques par une diminution de sa subvention pour charges de service public.

Il s’agit en effet de traiter cet opérateur sur un pied d’égalité avec les autres opérateurs de l’État au travers d’une diminution de 10 % de cette subvention, et non de 14 % comme le prévoyait initialement le projet de loi.

Sans renier notre objectif de redressement des finances publiques, nous devons préserver la capacité d’action de cet acteur important pour l’économie touristique de notre pays. Vous le savez, nous sommes dans une période de capitalisation sur les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) J’en viens maintenant aux enjeux en matière d’économie sociale, solidaire et responsable (ESSR), qui représente 14 % de l’emploi salarié, 10 % du PIB, plus de 155 000 entreprises employeuses et 22 millions de bénévoles.

Pour ce changement d’échelle, les politiques de soutien aux écosystèmes territoriaux, les dispositifs locaux d’accompagnement aux chambres régionales de l’ESS (Cress), notamment, sont indispensables. Aussi, afin de préserver les leviers d’action nécessaires au développement de l’économie sociale et solidaire dans tous les territoires, le Gouvernement présentera un amendement visant à rehausser les crédits en faveur de l’ESSR de 10 millions d’euros,

à une subvention de fonctionnement et d’investissement. Il est logique que ces dépenses ne soient pas reconduites cette année, ce qui ramène le financement à l’unique subvention pour charges de service public à hauteur de 42,5 millions d’euros. La DGCCRF continuera en 2025 d’être mobilisée sur les questions de relations commerciales. Plus largement, ses actions en matière de loyauté des transactions – informations relatives aux prix, licéité des contrats et des ventes promotionnelles – concourront à limiter le poids du contexte économique sur les consommateurs les plus exposés. La protection du consommateur sur internet se traduira notamment par le renforcement des contrôles des pratiques commerciales des influenceurs, des sites de livraison directe, de la mode éphémère ou de produits présentant un réel danger. Afin de soutenir la DGCCRF dans la mise en œuvre de ses missions, le Gouvernement propose un amendement visant à abonder les crédits

service d’un projet de décarbonation dans l’industrie est supérieur à trois ans. Il importe donc de donner de la visibilité aux porteurs de projets dès à présent, afin de sécuriser la mise en service de projets à moyen terme. Le soutien public octroyé à la décarbonation de l’industrie est une dépense efficace, dont le

développement d’une filière de production française de carburants aéronautiques durables, dans le cadre de la stratégie nationale « Produits biosourcés et biotechnologies industrielles Carburants durables de France 2030. Ces fonds permettent notamment de soutenir financièrement des projets de démonstration de procédés de production de carburants aéronautiques durables et des travaux de pré ingénierie de processus nécessaires pour engager un projet de production

L’Arcep a évalué à 322 millions d’euros le coût

l’avis de la commission ? D’assez nombreux amendements visent à augmenter la compensation versée par l’État au groupe La Poste au titre de ses missions de service public d’aménagement du territoire. La question de la sous compensation de cette mission de service public est un réel sujet et doit faire l’objet d’une réflexion plus large. Celle ci ne peut en effet pas être réglée par un simple amendement de crédits sur

revanche un avis favorable sur l’ensemble des amendements identiques à ceux de la commission et du Gouvernement, qui visent à porter le niveau de compensation pour 2025 à celui qui est prévu dans le contrat signé entre La Poste et l’État.

Cela nous paraît une position équilibrée. Il semble par ailleurs, madame la ministre, et je rejoins les propos de M. Chaize, que le PLFG pour 2024 prévoie de rétablir 35 millions d’euros sur les 50 millions

et près de 1 500 structures. Cette filière répond à un double objectif : c’est une économie à la fois prospère et sociale. Il ne s’agit pas d’une démarche philanthropique ou d’une béquille d’un régime socio économique en crise. Elle constitue une alternative enviable qui doit recueillir toute l’attention des pouvoirs publics.

Elles soutiennent la montée en compétence, la structuration et l’accès aux marchés publics des entreprises de l’ESS. La réduction des crédits prévue dans le PLF pour 2025 affaiblit leur capacité à répondre aux défis écologiques et sociaux auxquels nous faisons face. Avec cette augmentation, je souhaite renforcer leurs missions d’accompagnement et garantir qu’elles puissent continuer à jouer leur rôle qui est indispensable. Quel

2 millions d’euros, pour démarrer ce fonds et donner les moyens financiers et techniques pour transformer le modèle économique de ces entreprises. La transition vers une économie plus durable ne peut pas reposer

et que cette perte d’effectifs constatée depuis 2007 est tout à fait préjudiciable. Par exemple, dans le cadre des lois Égalim, la DGCCRF doit veiller à la juste rémunération des producteurs et au respect des modalités fixées

nécessaire à notre pays. Le lancement en 2021 du plan France 2030, doté de 54 milliards d’euros, a suscité de l’espoir, notamment auprès des acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui pensaient pouvoir en bénéficier. Alors que les acteurs de la transformation écologique et sociale ont besoin de moyens financiers pour se développer, l’innovation sociale et écologique est aujourd’hui sous financée. En témoignent les crédits fléchés dans la mission France 2030 100 % des investissements de la mission concernent des innovations technologiques –, ainsi que le sous subventionnement du secteur de l’ESS en France – une baisse de 25 % des financements est prévue par rapport à 2024. nous savons que la transition écologique ne pourra pas advenir sans un soutien aux transformations dans les usages des biens et services. Ces transformations d’usage, des innovations sociales et écologiques, ne naissent pas spontanément. Elles demandent des efforts de recherche et développement, puis d’industrialisation. Elles suivent les mêmes cycles économiques que les innovations technologiques, de l’investissement à l’exploitation. Afin de construire un plan de financement massif de l’innovation sociale et écologique, l’association Opération Milliard a réuni des milliers de dirigeants d’organisations d’innovation sociale de toutes formes économiques – sociétés de capitaux, coopératives, associations. Elle a permis qu’ils s’accordent sur une vision de la transition écologique juste et sur des modalités de financement de leurs actions afin de passer à l’échelle. Pour cela, ces organisations ont besoin de lever 1 milliard d’euros. Le soutien citoyen, mais aussi bancaire et public sera indispensable à la mise en œuvre de l’opération. L’État doit s’engager plus fortement pour soutenir les innovations sociales et écologiques nécessaires à la transition. Il peut, à travers l’augmentation du budget consacré à l’ESS au sein du programme 305 « Stratégies économiques », structurer une filière d’avenir et faire de la France un champion international de l’innovation sociale à dimension écologique.

En effet, alors que les entreprises bénéficient de mesures fiscales pour financer leurs programmes de recherche et d’innovation, les organismes sans but lucratif ne bénéficient pas de soutien au titre de leurs actions d’innovation sociale. Il est rappelé que l’innovation sociale a été définie légalement : est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant certaines caractéristiques caractéristiques – soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les organismes sans but lucratif sont confrontés à de nombreux défis – déserts médicaux, vieillissement de la population, cumul des freins sociaux des bénéficiaires, etc. – qui les obligent à innover socialement, en créant de nouveaux services et de nouvelles méthodes au plus proche des besoins des personnes accompagnées et de leurs familles. Cela implique des dépenses nouvelles, aussi bien en termes d’investissement en matériels et en équipements, que de fonctionnement – recrutement et formation du personnel. Ces investissements innovants comprennent souvent le recrutement de salariés, dont les salaires ne peuvent pas être financés par les ressources propres des structures. L’organisme sans but lucratif doit donc chercher des financements alternatifs, sous forme de don ou de mécénat par exemple. En outre, ses salaires sont soumis à la taxe sur les salaires. L’absence de financement public et l’assujettissement à la taxe sur les salaires sont des freins importants à l’innovation sociale. De toute évidence, il manque un soutien financier pour les organismes non soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun pour valoriser la recherche et soutenir l’innovation sociale qu’ils développent. Ce soutien en faveur de l’innovation sociale dans le secteur non lucratif pourrait prendre la forme d’une prime à l’innovation sociale à destination de ces organismes, dotée d’une enveloppe de 200 millions d’euros. Ce chèque représenterait environ 10 % des rémunérations brutes des salariés des entreprises de l’économie sociale et solidaire affectés aux projets d’innovation sociale.

aux entreprises de Bpifrance, de son activité d’accompagnement et de sa contribution au plan Quartiers 2030. La suppression des crédits affectés à Bpifrance actuellement prévue dans le PLF pour 2025 serait en effet lourde de conséquences. Compte tenu de l’efficience de ce plan et de son impact, il convient de pérenniser l’action de

ces amendements sur la nécessité pour le Parlement de disposer d’un contrôle sur les financements accordés à Bpifrance. Nous nous étions félicités, lors de l’examen du PLF pour 2024, de la création d’une ligne budgétaire dédiée au sein du programme 134.

adapter sa trajectoire financière au regard des contraintes budgétaires qui pèsent sur nous. Le Gouvernement soutient l’autofinancement par Bpifrance des dispositifs d’accompagnement et du plan entrepreneurial Quartier 2030. Bpifrance peut et doit trouver les capacités en interne compte tenu de son niveau de ressources propres, qui est aujourd’hui significatif.

» doté de 60 millions d’euros afin d’assurer le financement de CCI France et CMA France, en compensant la baisse du plafond des taxes affectées prévue par le PLF pour 2025. Cette baisse du plafond contrevient à la trajectoire financière pluriannuelle définie par le Gouvernement, le Parlement et le réseau des chambres de commerce et

notamment en matière d’inclusion numérique. Cette mission est particulièrement cruciale dans les zones rurales, où les enjeux de mobilité et l’éloignement des services publics renforcent les inégalités. Il est donc important de maintenir les engagements budgétaires dans ce domaine.

pouvoir les utiliser pleinement. Ces conseillers numériques jouent donc un rôle essentiel dans l’accompagnement de tous les citoyens et citoyennes vers l’inclusion numérique, sociale, professionnelle, culturelle, démocratique et citoyenne. Maintenir ces crédits, c’est lutter contre la progression d’une France à deux vitesses : celle des inclus et celle des exclus. La parole est à M. Damien Michallet,

des financements accordés aux conseillers numériques. Les crédits baissent de 33 % alors que les besoins persistent et que la fracture numérique est loin d’être résorbée dans notre pays. La commission des finances demande toutefois

locales, ces crédits ayant vocation à financer des dépenses engagées sur plusieurs années. Par ailleurs, cette situation entame la confiance des acteurs locaux, dans un contexte délicat de fermeture programmée du réseau de cuivre. Pour éviter une année blanche et soutenir les élus les plus en difficulté, nous proposons donc un rehaussement de 50 millions d’euros

les crédits de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » demandés pour 2025 s’élèvent à 21,5 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 21,6 milliards d’euros en crédits de paiement,

Pour autant, l’ampleur exacte de cette contribution n’est pas aisée à appréhender. En effet, la mission « Travail et emploi » du PLF pour 2024 est devenue la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux », en raison d’une modification de son périmètre. Elle s’est ainsi vu transférer les crédits support de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » et le programme 155, qui constitue le programme support de notre mission, a vu ses crédits multipliés par presque trois. Pour prendre la véritable mesure de la diminution des crédits de la mission par rapport à la loi de finances initiale pour 2024, il convient donc de raisonner à périmètre constant. Ce faisant,

Je le dis au cas où certains auraient des amis qui seraient tentés de ne pas voter le budget de cette année et, par voie de conséquence, Comme les années précédentes, l’évolution des dépenses de la mission dépend largement de celle des crédits du programme 103. En effet, celui ci participe pour une grande part au financement de l’apprentissage, qui constitue sa politique phare. Si on prend en compte l’ensemble des dépenses en faveur de la formation en alternance – les aides aux employeurs d’apprentis, les exonérations de cotisations en faveur de l’apprentissage et la dotation de l’État à France Compétences –, les crédits dédiés à cette politique sur le budget de l’État s’établissent à 7 milliards d’euros. Si on élargit encore la focale, et que l’on s’intéresse au coût de l’apprentissage pour l’ensemble des finances publiques, on prend conscience que celui ci est extrêmement important.

Le Gouvernement semble du même avis, puisque le PLF pour 2025 intègre une diminution de 663 millions d’euros en autorisations d’engagement des crédits dédiés aux aides aux employeurs d’apprentis. traduit sa volonté de réaliser une économie de 1,2 milliard d’euros par rapport à l’évolution tendancielle de ces dépenses. Toutefois, les modalités permettant de parvenir à ce résultat ne sont pas encore arbitrées.

qu’une mesure de ciblage devrait être prioritairement retenue plutôt qu’une baisse de la prime, mais nous n’excluons pas une solution qui allierait les deux. Nous sommes parfaitement ouverts à la discussion. La commission a également adopté un amendement pour tirer les conséquences de ce ciblage des aides sur les crédits de la mission. En conclusion, je dirai un mot sur l’esprit dans lequel la commission a examiné les amendements dont nous nous apprêtons à débattre nous pensons que l’état des finances publiques de notre pays exige des efforts importants, en particulier de cette mission budgétaire, dont les crédits ont fortement augmenté au cours des dernières années.

j’abonde dans le sens d’Emmanuel Capus. Ce n’est pas tous les jours, donc qu’il en profite… Depuis 2020, l’introduction de la prime dite exceptionnelle à l’embauche d’une personne en apprentissage a conduit à la hausse considérable du nombre d’apprentis. Cette aide, destinée aux employeurs, n’est pas ciblée et fonctionne en guichet ouvert, c’est à dire qu’elle est accessible sans limite à tous les candidats éligibles qui y postulent et en remplissent les conditions. Toutefois, la commission des finances du Sénat considère que le versement d’une telle aide présente un risque élevé d’effet d’aubaine.

Maintenir cette politique d’apprentissage en l’état pour 2025 serait disproportionné au regard du niveau de déficit de notre pays. C’est pourquoi nous vous proposons ce recentrage en faveur des petites entreprises et des jeunes les moins qualifiés. Dans la même veine, la commission des finances avance une autre piste d’économies, inspirée des recommandations de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection des affaires sociales (Igas) : celles ci préconisent de reconsidérer la prise en charge des coûts pédagogiques des contrats d’apprentissage, financés par France Compétences au niveau de prise en charge (NPEC) fixé par les branches professionnelles. Les inspections ont en effet mis en évidence le coût comparativement plus élevé des formations de niveaux licence et master. Conformément à ces recommandations et compte tenu de notre volonté de cibler le soutien public à l’apprentissage vers les niveaux de qualification pour lesquels ce soutien est le plus déterminant, nous vous proposons un amendement visant à limiter le financement des NPEC

J’insiste de nouveau sur le fait que nous avons souhaité engager un dialogue avec le Gouvernement, qui a lui même déposé un amendement visant à diminuer les crédits de la mission de 675 millions d’euros supplémentaires. Autant le dire franchement,

qui entraînerait des restrictions sur les divers dispositifs favorisant l’accès à l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées. On ne peut pas, d’un côté, consacrer des dizaines de milliards d’euros à l’insertion professionnelle des diplômés du supérieur, souvent des cadres – 61 % des bénéficiaires de l’apprentissage proviennent des formations de l’enseignement supérieur

La commission se prononce favorablement sur la suppression des contrats aidés dans le secteur marchand, ainsi que sur celle des emplois francs, arguant que la légitimité de ces dispositifs peut être remise en cause par les effets d’aubaine très importants qu’ils suscitent. Pour ma part, je ne partage pas tout à fait cet avis. Je m’inquiète par ailleurs de la diminution des crédits dédiés aux missions locales. En effet, les crédits de paiement qui leur seraient alloués baisseraient de 22,2 % entre la loi de finances 2024 et le présent PLF.

Je souhaite aussi dire quelques mots de la dette de l’Unédic, qui est estimée à 58,4 milliards d’euros fin 2024. Depuis 2023, l’État ponctionne une partie des excédents de l’association : 2 milliards d’euros en 2023, 2,6 milliards en 2024 et 3,35 milliards prévus en 2025. Ces ponctions ralentissent la trajectoire de désendettement de l’Unédic, ce qui n’est pas anecdotique, compte tenu du rôle de stabilisateur automatique de l’assurance chômage. Nous risquons d’entrer dans un cercle vicieux extrêmement défavorable. Enfin, je veux attirer votre attention, mes chers collègues, sur la situation des acteurs de l’insertion par l’activité économique Si leurs moyens sont globalement préservés, nous avons été alertés sur le fait qu’ils pourraient être insuffisants pour absorber la hausse prévue du Smic et maintenir les effectifs à leur niveau de 2024. Bien que la commission ait rendu des avis globalement défavorables sur les amendements visant à revenir sur les baisses de crédits que je viens de désigner, je vous indique que je suis, à titre personnel, favorable à ces initiatives.

Cette baisse de la dépense publique a beau être l’une des principales du budget de l’État cette année, gardons toutefois à l’esprit que les crédits demandés restent toujours supérieurs de plus de 6 milliards d’euros par rapport à ceux La commission des affaires sociales a soutenu la diminution proposée, à l’aune de trois objectifs : placer les dépenses de cette mission sur une trajectoire soutenable sur le long terme ; porter une attention à la qualité des dispositifs financés ; veiller à ne pas sacrifier l’application de réformes structurelles importantes. Dans ce contexte, notre commission a d’abord considéré que les moyens alloués au service public de l’emploi, et notamment à France Travail, ne devaient pas mettre en péril la mise en œuvre de loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, texte rapporté Nous prenons ainsi acte de la stabilité de la subvention accordée à France Travail, conformément à la trajectoire prévue par la convention tripartite conclue le 30 avril 2024. Toutefois, la diminution de ses effectifs de 500 ETP demandée à l’opérateur ne nous paraît pas prendre en compte les besoins réels induits par loi précitée.

la commission des lois pour les crédits du programme 148 « Fonction publique ». Concernant les crédits alloués à la formation professionnelle, il nous paraît nécessaire de soutenir la maîtrise des dépenses d’alternance. Toutefois, la commission estime que cette régulation doit s’engager sans casser la dynamique de l’apprentissage et sans risquer une détérioration de l’accompagnement des apprentis. Le PLF est construit sur l’hypothèse d’une aide aux employeurs d’apprentis abaissée uniformément à 4 500 euros, contre 6 000 euros actuellement. Nous pensons que cette diminution peut être trop brutale, à plus forte raison pour les TPE et les PME. Nous proposerons donc de porter ce montant à 5 000 euros. En revanche, comme le propose la commission des finances, cette aide ne serait plus versée pour les niveaux de qualification bac+3 et au delà dans les entreprises de plus de 250 salariés. Enfin, nous avons été attentifs à l’équilibre budgétaire de France Compétences. Son déficit prévisionnel, qui s’élève à 464 millions d’euros pour 2025, montre que, cette année encore, le financement de l’apprentissage n’est pas assuré. Cet équilibre est pourtant atteignable et la commission propose deux mesures à cette fin. D’une part, nous estimons que la contribution de France Compétences au plan d’investissement dans les compétences (PIC) n’est pas souhaitable, alors que le financement des missions premières de l’opérateur n’est toujours pas assuré.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » du projet de loi de finances est sans doute l’une des plus importantes pour nos concitoyens. Avec des crédits en baisse de 10,2 % par rapport à 2024, elle aussi l’une de celles qui subissent le plus l’effort de réduction des dépenses de l’État demandé pour 2025. Si le groupe RDPI consent à cet effort nécessaire au redressement de nos comptes publics, il estime que ledit effort ne doit pas se faire au détriment des résultats obtenus depuis 2017, notamment dans la recherche du plein emploi. Nous partageons toutefois les grands objectifs affichés dans le PLF pour cette mission. L’année 2025 verra se poursuivre le déploiement de France Travail, la mise en œuvre de mesures dans les champs de l’emploi et de la formation des jeunes, ainsi que l’amélioration des conditions de travail et de la santé au travail. Les principales mesures de la réforme de l’accompagnement des demandeurs d’emploi doivent entrer en vigueur au 1 janvier 2025. Il s’agit en particulier de l’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi de France Travail de toutes les personnes éloignées de l’emploi. Nous souscrivons aussi au renforcement de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans le cadre du contrat d’engagement unifié. 2025 prévoit de maintenir à 1,35 milliard d’euros la subvention de l’État à l’opérateur France Travail, afin de poursuivre le déploiement de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi ; nous soutenons cette

cadre du contrat d’engagement prévu par la loi pour le plein emploi et ses bénéficiaires seront inscrits en tant que demandeurs d’emploi à France Travail. Le PLF pour 2025 prévoit une stabilité des crédits de financement des CEJ et nous nous en réjouissons. Parce qu’il ne faut laisser personne au bord du chemin de l’insertion professionnelle, il nous faut aussi continuer de soutenir le secteur de l’insertion par l’activité économique et les aides au poste dans les entreprises adaptées ce PLF est assez ambitieux en la matière. Évoquons maintenant le sujet de l’apprentissage. Nous l’avons dit lors de la discussion du PLFSS, il est hors de question pour notre groupe de sacrifier cette politique conduite avec succès depuis 2017 sur l’autel de la situation budgétaire.

Dans certains secteurs, freiner brutalement l’apprentissage pourrait mettre à mal une voie historique de formation aux métiers. Nous serons attentifs à ce que des critères justes soient définis, tant pour réduire les effets d’aubaine que pour pérenniser le soutien apporté

l’équilibre est atteignable en 2025 grâce à la mise en extinction du financement du PIC par l’opérateur, combinée à la suppression de l’éligibilité de droit au CPF des actions de formation pour la création ou la reprise d’entreprise, qui fait l’objet d’abus. Il nous faudra aussi continuer à défendre un dialogue social exigeant et de qualité, malgré une diminution des crédits alloués à ce programme. Nous approuvons par ailleurs le financement à hauteur de 1 million d’euros du soutien à la révision ou à la refonte des systèmes de classification des branches professionnelles.

dont l’expérimentation n’a pas encore démontré la pleine efficacité. Il faudra enfin veiller à la bonne adaptation de cette mission à la spécificité des outre mer – j’y tiens tout particulièrement. Madame la ministre, malgré quelques divergences, notre groupe votera cette mission et nous comptons sur vous pour tenir le

de seniors au chômage, parmi lesquels on retrouve beaucoup de femmes. Il y a également toujours plus d’actifs occupant des contrats courts et toujours plus de précarité parmi les jeunes peu qualifiés, qualifiés ou issus de milieux modestes.

Soucieux d’une meilleure prise en charge de ces publics, et en particulier des générations qui entrent sur le marché du travail, notre groupe a déposé plusieurs amendements visant à élever notre niveau d’ambition en matière d’apprentissage et d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Philippe Grosvalet, notre attachement aux missions locales, qui constituent le premier réseau de service public pour l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans vers l’insertion sociale et professionnelle. Les défis relevés par les missions locales sont si grands et si rudes qu’il convient de leur octroyer des moyens adaptés, qui plus est lorsqu’elles subissent déjà des baisses de subventions de la part de certaines collectivités territoriales. Par ailleurs, notre collègue Véronique Guillotin, élue de Meurthe et Moselle, département où vivent de nombreux travailleurs frontaliers, a légitimement souhaité déposer un amendement sur le système d’indemnisation des allocataires frontaliers dans le cadre de l’assurance chômage. Vous le savez, c’est un problème qui coûte à l’État environ 800 millions d’euros par an et qui préoccupe grandement les travailleurs concernés. Il devient urgent d’engager des négociations avec les États voisins afin de conclure des accords bilatéraux plus justes au regard des réalités économiques. À nos yeux, l’expertise locale de proximité doit rester au cœur des politiques de l’emploi. Nous comptons à cet égard sur le rôle pivot des opérateurs historiques, mais aussi sur les régions, les départements et les communes.

être atteints. Parce que le travail conditionne l’émancipation des individus, la cohésion sociale, mais aussi la dynamique de l’économie française, la responsabilité des pouvoirs publics dans ce domaine est essentielle.

dans ce contexte financier, social et politique extrêmement tendu, il est de notre responsabilité de proposer des mesures fortes afin de rééquilibrer les comptes publics, mais nous ne devons pas pour autant déstabiliser notre économie. Les enjeux sont grands : comment fidéliser les employés dans certaines filières et pérenniser des postes dans d’autres ? Nous, centristes, appelons à la mesure et à l’équilibre, car nous sommes sur une ligne de crête

Accordons leur un financement adapté aux missions qui leur ont été confiées par la loi pour le plein emploi, car leurs contraintes sont multiples : infrastructures insuffisantes pour accueillir des ateliers,

viens maintenant au financement de l’apprentissage. La commission des affaires sociales a appelé le Gouvernement à faire preuve de vigilance afin que la diminution du financement de l’apprentissage ne soit pas trop brutale. Il faut de la mesure et du pragmatisme pour continuer à développer une politique ambitieuse

l’idée centrale étant : aider moins, oui, mais aider mieux, assurément ! Nous devons éviter le raccourci suivant : les petites entreprises embaucheraient à de petits niveaux de diplômes. Leur besoin d’apprentis à haut niveau de qualification est bien réel : ne nous méprenons pas L’apprentissage participe au bon fonctionnement de l’ascenseur social et correspond à une demande des entreprises, celle de former des travailleurs qualifiés, qui sont nécessaires à la pérennité de leurs activités. Préservons l’apprentissage, qui est devenu une filière d’insertion reconnue, une formation d’excellence pour les jeunes à tout niveau de qualification, et un investissement sur l’avenir pour les entreprises. Réduire les dépenses est est une nécessité budgétaire, mais porter atteinte à l’emploi et à l’insertion professionnelle des jeunes, je ne peux m’y résoudre ! La parole

Tout au long de l’examen du PLFSS et de la première partie du PLF, nous avons proposé des recettes nouvelles : taxer les dividendes, conditionner les aides publiques aux entreprises, revenir sur les exonérations de cotisations. Par choix dogmatique, vous avez refusé de taxer les plus riches et décidé de faire payer les ouvriers et les familles les plus fragiles. L’examen des crédits de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux » s’inscrit dans un contexte particulièrement lourd pour l’emploi dans notre pays. Selon la CGT, près de 250 plans de licenciement sont en préparation dans l’industrie, soit 200 000 emplois menacés dans les prochaines semaines. Chaque emploi supprimé entraîne un effet domino sur les sous traitants, sur les prestataires de services et sur tout l’écosystème économique local. Ces plans de licenciement n’effacent pas seulement des emplois, ils privent des régions de leur attractivité et les vident de leurs commerces de proximité. Ce sont des vies brisées, des familles dans l’incertitude : derrière les chiffres, c’est un drame humain qui se joue et le Gouvernement n’anticipe rien. La CGT sonne l’alarme pour éviter l’érosion de notre industrie, déjà fortement minée par trente ans de libéralisation et de concurrence européenne. Les salariés sont appelés à faire grève le 12 décembre et à occuper leurs usines pour empêcher les licenciements ; nous serons à leurs côtés face à l’abandon des gouvernements successifs. Les entreprises qui ont été gavées d’aides publiques rechignent aujourd’hui à abandonner une part symbolique des 250 milliards d’aides annuelles. Les mêmes qui ont imposé des conditions draconiennes aux travailleurs et aux allocataires du RSA pour qu’ils puissent bénéficier de leurs droits estiment qu’il serait inconcevable que les entreprises s’engagent à mieux rémunérer leurs salariés, à respecter l’égalité salariale ou à mieux prendre en considération l’environnement en contrepartie des milliards distribués chaque année.

réduction des dépenses touche les dispositifs d’accompagnement des plus fragiles, avec une baisse des moyens alloués à l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi et une baisse de 10 % des crédits destinés à l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Les réductions concernent également les moyens de la formation continue et de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi. C’est un coup de massue pour un public souvent en reconversion ou non diplômé. La baisse des crédits dévolus aux structures de la formation professionnelle et de l’emploi pour 2025 s’inscrit par ailleurs dans une trajectoire de réduction des moyens qui dure depuis plusieurs années et met en danger la pérennité de certains établissements comme l’Agence Comme un symbole de la politique du Gouvernement, le programme « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » voit ses crédits diminuer de 24 %, soit une baisse de 30 millions d’euros par rapport à 2024.

et, surtout, des médecins du travail. Le Gouvernement trouve encore l’occasion de réduire les crédits pour le dialogue social et la démocratie sociale de 32 %, alors même qu’ont déjà été supprimés les

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après sept années d’impéritie budgétaire qui ont grevé les recettes et créé des déficits, lesquels ont ensuite justifié des contre réformes systémiques injustes, le Gouvernement présente un budget austéritaire, dont le principal credo est est le coup de rabot sur les dépenses publiques, sans jamais interroger ses choix politiques inconséquents. Pourtant, à lire les derniers rapports de la Cour des comptes, il est aisé de constater

t elle que la « période 2018 2023 a été marquée par d’importantes baisses d’impôts, dont l’impact est [de] 2,2 points de PIB », précisant que ce sont bien les « baisses de prélèvements obligatoires mises en œuvre à partir de 2018 » qui ont provoqué une grande partie du déficit. Or, au lieu de revenir, du moins en partie, sur cette politique d’attrition des recettes de niches fiscales aux effets quasi nuls sur l’emploi et la compétitivité, mais aux coûts croissants, le Gouvernement comble le déficit un budget austéritaire, dont l’effet récessif pour l’année 2025 a été estimé à 0,8 point de PIB par l’OFCE.

des accidents et des morts au travail. On note également une fragilisation des structures d’insertion, quel que soit le modèle, des entreprises d’insertion aux chantiers d’insertion, ainsi que la non revalorisation le gel – des aides au poste, dans un contexte où un tiers des entreprises d’insertion et la moitié des chantiers d’insertion sont en difficulté financière.

Toutes ces mesures austéritaires antisociales sont à contretemps du contexte social et économique : l’OFCE prévoit un retournement de la conjoncture et une augmentation du chômage en 2025, et les défaillances et les plans sociaux se multiplient. mesures vont surtout à rebours de la loi Plein Emploi : la stagnation des crédits alloués à France Travail et les difficultés des structures d’insertion conduisent à un véritable sabordage des maigres

l’aveugle 500 postes, mesure insuffisamment corrigée par la commission des affaires sociales du Sénat. En réalité, le Gouvernement condamne sa propre réforme à l’échec et renvoie les dépenses sur les départements, dont il contraint par ailleurs le budget. Il ne peut ignorer que cette politique dopera l’externalisation des missions publiques vers des opérateurs privés de placement, dont l’efficacité est moindre pour un coût deux fois plus élevé. Désormais, le seul credo est la rigueur budgétaire, et ce pour ne pas toucher aux niches fiscales et sociales. Tant pis si ce plan d’ajustement structurel mène à la précarisation du travail, au renforcement de l’exclusion sociale et à l’affaiblissement des moyens de l’État ! Mieux vaut lorgner les excédents de l’Agirc Arrco, faire les poches de l’Unédic en déstabilisant sa trajectoire budgétaire

Pendant sept ans, l’exécutif a balayé les propositions politiques des oppositions en se prévalant d’être l’unique option responsable. Le résultat, c’est un déficit historique et un nombre record de personnes en

la centralité du travail pour notre insertion dans la société, le sens que nous y mettons, la manière dont les droits des individus en emploi sont respectés, la place de la valeur travail et la manière dont nous réussissons collectivement à prendre en charge ces enjeux : c’est notamment de ces sujets que traite la mission

La revendication d’une efficacité accrue du « faire plus avec moins » fait office d’illusoire principe directeur. L’art de créer des tuyaux pour ponctionner certains budgets, pendant qu’une diversion s’opère au moyen d’un saupoudrage de moyens cosmétiques sur d’autres secteurs, est encore une fois à l’œuvre ici. Les véhicules législatifs qui permettent ce jeu de bonneteau sont notamment la loi pour le plein emploi et les projets de loi de finances successifs. Le programme 102 « Accès et retour à l’emploi » nous interpelle notamment en ce qui concerne le sort qui y est réservé à France Travail. Pour mémoire, la loi pour le plein emploi réforme l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, en prévoyant notamment leur inscription automatique à France Travail. Cela représente une importante charge de travail supplémentaire.

au risque de déposséder les acteurs locaux (missions locales, départements, travailleurs sociaux…) de leur savoir faire et de leurs moyens d’action et d’évaluation.

proposée par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi. La conclusion des chercheurs est sans équivoque : « La présente recherche met en exergue les atteintes psychiques provoquées par la confrontation à Pôle emploi. » Vu ses nouvelles missions, le service public de l’emploi ne peut de toute évidence pas se permettre une diminution de ses moyens humains et financiers. Dans ce contexte, la sous Dans ce contexte, la sous traitance par le Gouvernement des tâches de France Travail, récemment mise en avant par, est une forme d’inadmissible cerise sur le gâteau

Avec France Travail, une nouvelle externalisation massive est prévue. Un accompagnement dédié à la reprise rapide d’emploi va être sous traité à des opérateurs privés. C’est le parcours dit de reprise rapide d’emploi qui est en cause. Il devrait concerner de 700 000 à 900 000 privés d’emploi chaque année et aura un coût de 448 euros par usager Par ailleurs et en tout état de cause, la baisse du chômage dont les concepteurs de ce budget se prévalent pour justifier la baisse des moyens de France Travail est un argument inaudible. Dans une note du mois d’octobre 2024, l’OFCE prévoit ainsi que le chômage progresse d’au moins 0,5 point pour atteindre 8 % à la fin de l’année 2025. Ce sont 143 000 emplois qui devraient être détruits au cours de cette période. Toujours au titre du programme 102, le sort réservé aux missions locales et aux contrats aidés ne nous a pas échappé. des missions locales sont en forte diminution, ce à quoi nous nous opposons fermement – nous y reviendrons au cours de la discussion. Nous ne saurions accepter une telle diminution. Les crédits

se heurte aussi à l’absence d’alternative opérationnelle à ces contrats si le chômage remonte, car les publics fragiles à insérer en emploi sont alors plus nombreux. » La diminution du budget alloué aux contrats aidés est cohérente avec les arbitrages qui ont été faits ces dernières années par l’exécutif hormis pendant les périodes de crise, ce dernier a clairement tendu à couper dans les enveloppes consacrées auxdits contrats, et ce dès l’entrée en fonction d’Emmanuel Macron. Une étude de la Dares de 2017 soulignait pourtant leur efficacité. Les affaiblir est la marque d’une politique qui n’est ni visionnaire ni responsable. viens à l’insertion par l’activité économique, chère à nombre de mes collègues – je pense notamment à Patrice Joly, qui a tenu à m’informer de difficultés sur son territoire. Le montant affecté au financement direct de ce secteur pour 2025 reste à peu près constant par rapport à 2024. mes chers collègues, j’appelle votre attention sur les associations intermédiaires. Elles assument une mission de service public et sont un employeur d’insertion majeur. Le maillage territorial qu’elles tissent fait d’elles, bien souvent, les seules structures présentes dans les territoires économiquement Elles assument donc un rôle essentiel de créateur de lien social, d’accueil, d’écoute, d’accompagnement socioprofessionnel et d’orientation : autrement dit, elles assurent un quasi service public de l’emploi.

Les soutenir en ce moment, alors que les difficultés risquent de s’accentuer pour les personnes en recherche d’emploi, est plus que nécessaire. Elles ont en effet elles aussi affronté l’inflation, qui les a mises en grande difficulté.

dans le domaine de l’apprentissage nous laissent perplexes. Après l’avoir soutenu massivement en vue d’atteindre l’objectif du million d’apprentis, objectif qui n’a d’ailleurs pas été atteint, le Gouvernement prévoit une diminution de près de 50 000 contrats par rapport à 2024. De plus, l’enveloppe budgétaire globale pour 2025 baisse de 1,2 milliard d’euros par rapport à l’année précédente. Il est difficile de lire la politique du Gouvernement en la matière

la qualité du droit, sa diffusion et le contrôle de sa mise en œuvre, le conseil et l’appui au dialogue social. Les crédits de paiement alloués à ce programme sont de 83,6 millions d’euros en 2025, soit une baisse de 24 % par rapport à 2024. à 2024. À l’appui des propositions d’amendement que nous ferons dans ce champ, je rappelle par exemple que, chaque année, près d’un million d’accidents surviennent, dont plusieurs centaines sont mortels, et près de 50 000 nouvelles reconnaissances de maladies professionnelles sont comptabilisées. Le renforcement des droits des travailleurs, donc de l’inspection du travail, fait ainsi partie de nos préoccupations majeures.

de remanier en profondeur le budget de cette mission pour garantir à nos concitoyens l’accès au service public de l’emploi auquel ils ont droit. La parole est à M. Jean Luc Brault. Monsieur le président,

s’inquiéter serait être aveugle à l’état de santé de nos entreprises, petites ou grandes, et au quotidien de bon nombre de travailleurs et de compagnons, quels qu’ils soient, où qu’ils soient.

Soyons réalistes : au regard de la situation politique de notre pays, ce n’est pas fini ! Il nous faut regagner de la confiance dans notre économie. Je l’ai indiqué lors de l’examen de la mission « Économie », je le répète : il nous faut du courage, beaucoup de courage, pour diminuer nos dépenses

et qui sera pleinement mise en œuvre l’année prochaine. Un autre sujet me tient particulièrement à cœur, madame la ministre : c’est l’apprentissage. Entre le coût financé par l’État, de l’ordre de 7 milliards d’euros, les différentes exonérations sociales ou le soutien de France Compétences, le total des dépenses publiques en faveur de l’apprentissage représenterait environ 25 milliards d’euros. Soyons clairs : l’apprentissage est une force, il est même parfois vital pour notre économie, pour nos territoires et pour nos entreprises.

L’apprentissage, c’est l’équation parfaite du donnant donnant : il fait naître des vocations chez les apprentis et pourvoit nos entreprises de salariés opérationnels et déjà intégrés ; et, demain, ces compagnons pourront réaliser à leur tour le bel ouvrage. a connu une formidable évolution depuis 2018, passant de 320 000 contrats à 849 000 en 2023. Il n’est pas question de le sacrifier. Nous sommes passés d’une voie de garage à une voie royale : maintenons cette belle dynamique.

ce domaine : le n’est pas tenable. L’année dernière, déjà, nous alertions sur la nécessité d’un meilleur ciblage des aides aux entreprises embauchant un apprenti. Si le ciblage actuel, très large, a grandement contribué au succès du dispositif, il a aussi entraîné des effets d’aubaine.

ces amendements vise à réaliser une économie de l’ordre de 300 millions d’euros, en concentrant les aides sur les plus petites entreprises et sur les apprentis dont le niveau de qualification est inférieur à bac+3 ; c’est une mesure de bon sens. Le second amendement vise à réajuster une situation incohérente : alors que les formations de niveau 6 et 7 – licence, master et doctorat – ne représentent respectivement que 18 % et 17 % des contrats, elles pèsent pour 40 % et 32 % de la prise en charge par France Compétences.

les moyens demandés au titre des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle s’élèvent à 21,6 milliards d’euros pour 2025, ce qui représente, à périmètre constant, une baisse de 10,2 % par rapport à 2024. serait donc le premier à enrayer la hausse continue des crédits de cette mission, lesquels ont progressé de 14,2 milliards d’euros en 2019 à 22,6 milliards d’euros en loi de finances pour 2024. Cette trajectoire ne paraissait pas soutenable ; la maîtrise des dépenses est donc une bonne chose. Elle doit permettre une allocation plus efficiente des crédits budgétaires. À cet égard, la proposition de la rapporteure pour avis Frédérique Puissat de diminuer les crédits des opérateurs de l’État rattachés à cette mission est bienvenue. qui est des dispositifs financés, il convient bien entendu de garder à l’esprit l’objectif, qui est de tendre vers le plein emploi, et ainsi de ne pas couper à l’aveugle dans les financements. En ce qui concerne l’insertion professionnelle, le grand enjeu de 2025 sera la mise en œuvre de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi. Dès l’année prochaine, le contrat d’engagement doit être mis en œuvre pour toutes les personnes privées d’emploi, dont les bénéficiaires du RSA, dans tous les territoires. Les financements prévus en 2024 pour les départements et pour la subvention destinée à France Travail sont maintenus dans ce PLF. En revanche, concernant le plafond d’emplois de France Travail, il convient de ne pas placer l’opérateur dans une situation paradoxale en lui demandant de mettre en œuvre des mesures ambitieuses tout en lui retirant les moyens humains de le faire. Ainsi que l’a indiqué la rapporteure pour avis, la baisse des effectifs proposée dans le texte initial risque de remettre en cause certaines réformes structurelles du marché du travail. Or, dans un objectif d’efficience de la dépense publique, il ne paraît pas souhaitable de compromettre la mise en œuvre du renforcement des contrôles de la recherche effective d’emploi, ni celle de la lutte contre les comportements abusifs, ni celle de l’accompagnement de 200 000 bénéficiaires du RSA en application de la loi pour le plein emploi. D’autres dispositifs concourent à l’insertion par l’emploi. Le secteur de l’insertion par l’activité économique bénéficierait d’un financement stable, à hauteur de 1,5 milliard d’euros. Nous avons bien sûr conscience que l’absence de revalorisation des aides au poste en parallèle de celle du Smic conduit en réalité à demander un léger effort au secteur. Celui ci reste toutefois mesuré dans le contexte budgétaire difficile que nous connaissons, ce qui est plutôt satisfaisant. Je pense également aux aides au poste dans les entreprises adaptées, dont les financements progressent de 7 % par rapport à 2024. Cette consolidation des moyens en faveur de l’insertion des travailleurs en situation de handicap est un effort bienvenu. J’en viens désormais aux crédits alloués à la formation professionnelle et à l’apprentissage. Le projet de loi de finances prévoit de restreindre de 660 millions d’euros l’enveloppe consacrée aux aides aux employeurs d’apprentis. Nous soutenons le principe d’une modération de ces dépenses, alors que le succès indéniable de l’apprentissage s’est accompagné, nous le savons tous, d’un coût absolument démesuré pour les finances publiques. Toutefois, nous pensons qu’il ne faut pas restreindre brutalement l’aide aux employeurs, sous peine de mettre en danger l’apprentissage dans certains secteurs, notamment dans les TPE et les PME. loi de finances est construit sur l’hypothèse d’une aide de 4 500 euros, la position de la commission des affaires sociales paraît mesurée en ce qu’elle maintient l’aide à 5 000 euros pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, sans distinction du niveau de qualification de l’apprenti. En outre, la situation financière de France Compétences reste préoccupante. Son budget devrait être déficitaire de 1 milliard d’euros en 2024 et de 464 millions d’euros en 2025. Les déficits cumulés de l’opérateur depuis 2019 devraient donc s’élever à près de 11 milliards d’euros en 2025. Nous saluons les mesures prises par l’opérateur pour réguler les dépenses de prise en charge des contrats d’apprentissage

au titre du compte personnel de formation devraient être stabilisées en 2024, grâce à la participation obligatoire du bénéficiaire, finalement mise en œuvre par un décret du 29 avril 2024, et grâce à l’encadrement du financement des permis de conduire.

Nous soutenons l’amendement de la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales qui vise à supprimer cette éligibilité de droit des actions Acre. Ces dernières resteraient éligibles au CPF, mais seulement dans le cadre de formations certifiantes inscrites aux répertoires nationaux. Enfin, nous pensons qu’il faut recentrer les dépenses de France Compétences sur la prise en charge de l’apprentissage. Comme les années précédentes, il n’est pas souhaitable que l’établissement participe au financement du plan d’investissement dans les compétences, le PIC. En outre, les mêmes incertitudes sur les objectifs et le pilotage du PIC demeurent cette année.

sous réserve de l’adoption des amendements de la commission des finances sur le financement des formations dispensées par les CFA et des amendements de la commission des affaires sociales. La parole

avant d’entrer dans le détail de la mission qui nous occupe, permettez moi de commencer mon propos, puisque nous parlons d’emploi, en rappelant que la France connaît 3 600 pertes d’emplois par semaine dans les entreprises, toutes tailles confondues, dont 1 219 dans les très petites Ces emplois passent sous les radars parce qu’ils ne sont pas forcément le fruit de grands plans de licenciement. Je souhaite également mettre l’accent sur la situation de la centrale thermique de Provence, à Gardanne dans les Bouches du Rhône. J’ose espérer, madame la ministre, qu’aucun ministère – je pense notamment à Bercy – ne reviendra sur sa parole et que les 500 emplois menacés seront sauvés comme annoncé, avant qu’une possible censure ne vienne remettre en cause les arbitrages actés par l’État. Aujourd’hui, la situation est inquiétante, et nous devons exprimer ici, au Sénat, notre désapprobation quant aux menaces qui pèsent sur le Gouvernement, et donc, en bout de chaîne, sur le monde du travail,

Concernant France Travail, ensuite, nous constatons là aussi une baisse des moyens alloués à cette structure la diminution des crédits aux opérateurs. Pour autant, les moyens mobilisés demeurent nettement supérieurs à ceux d’avant la crise sanitaire, et la subvention pour charges de service public, elle, est préservée.

Les 500 équivalents temps plein qui seront supprimés en 2025 constituent un ajustement budgétaire significatif. Je soutiens, comme la commission des affaires sociales, que la rationalisation des effectifs est compréhensible dans un contexte de maîtrise des finances publiques. Néanmoins, il est essentiel que cette réduction soit soigneusement calibrée pour ne pas compromettre l’application de réformes structurelles telles que le contrat d’engagement unifié, la généralisation du dispositif Avenir Pro ou le renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et des jeunes en CEJ. façon, la prospection des entreprises ne doit pas être mise en péril par une diminution aveugle des ressources humaines. Dans cet esprit, l’amendement visant à limiter la réduction à 205 postes est un compromis

parfois très élevé, doivent être répertoriées, analysées et, dans certains cas, lorsque cela se justifie, écartées. Pour conclure, je rappelle que la question de l’emploi pourrait être fortement bousculée dans les prochaines heures. Soyons responsables ! Le groupe Union Centriste, lui, prend ses responsabilités ; il votera pour cette mission. La parole

Ces crédits devraient toutefois permettre de concrétiser des mesures soutenues depuis longtemps au Sénat, comme le renforcement de l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans le cadre du contrat d’engagement unifié, les quinze heures d’activité exigées en contrepartie du RSA, ou encore la lutte contre les comportements abusifs. des affaires sociales de l’amendement de la rapporteure pour avis visant à augmenter le plafond d’emplois demandé pour France Travail. En effet, la contraction prévue dans la version initiale du PLF aurait risqué de mettre en péril des mesures importantes, comme la généralisation du dispositif qui permet enfin au réseau pour l’emploi de « sortir de ses murs » et de nouer un contact privilégié avec les entreprises. Cet amendement est également indispensable pour tenir l’objectif d’accompagnement de 200 000 bénéficiaires du RSA.

professionnels ou socioprofessionnels, on peut dire que cette expérimentation est un succès : à la clé, un meilleur accompagnement des bénéficiaires du RSA et davantage de solutions d’insertion pour favoriser leur retour à l’emploi. Saluons aussi le maintien par la commission des crédits au bénéfice des maisons de l’emploi à hauteur de 5 millions d’euros, afin de financer leurs fonctions socles d’ingénierie territoriale et de réussir leur intégration au sein du réseau pour l’emploi. est des missions locales, qui constituent le premier réseau de service public pour l’accompagnement des jeunes vers l’insertion sociale et professionnelle, il faudra veiller à ce que la réduction des crédits de 140 millions d’euros cible réellement certaines missions locales dont la trésorerie est excédentaire, comme l’a indiqué la Par ailleurs, j’encourage la labellisation des missions locales pour une meilleure organisation. En ce qui concerne les contrats aidés, le PLF pour 2025 prévoit une nouvelle baisse des crédits de 164 millions d’euros, ce qui se traduirait par une limitation à 50 000 du nombre de nouvelles entrées en parcours emploi compétences (PEC),

Or, dans certains secteurs, freiner brutalement l’apprentissage risquerait de mettre à mal une voie historique de formation aux métiers. C’est pourquoi je salue, là encore, l’amendement adopté en commission des affaires sociales qui vise à augmenter de 320 millions d’euros la ligne budgétaire attribuée à l’aide aux employeurs. aide ne s’appliquerait pas aux niveaux de formation égaux ou supérieurs à bac+3 dans les entreprises de plus de 250 salariés. L’adoption de cet amendement permettrait de ne pas casser la bonne dynamique de l’apprentissage tout en organisant un meilleur ciblage du soutien public à cette politique. Enfin, il est nécessaire de créer les conditions de l’équilibre budgétaire de France Compétences. Malgré les réductions inscrites dans le PLF, le budget de l’organisme devrait rester déficitaire de 464 millions d’euros

un meilleur emploi des moyens de France Compétences devra donc être l’une des priorités du Gouvernement, sans que soient fermés les petits CFA, si indispensables pour notre ruralité.

beaucoup de choses ont été dites par les rapporteurs et par les représentants des groupes. Je vais aller à l’essentiel, dire quelle est la cohérence de ce budget et répondre à certaines interrogations avant que nous n’entamions la discussion des amendements.

baisse des crédits. Cette diminution prolonge un exercice budgétaire 2024 au cours duquel, déjà, les crédits du ministère du travail ont été diminués de 1,1 milliard d’euros, en application du décret d’annulation du 21 février 2024. La contribution du ministère du travail a ainsi représenté plus de 10 % des annulations totales. Ces baisses sont importantes, chacun le reconnaît, moi la première. la première. Je tiens à vous rappeler quel est mon état d’esprit. Dans un cadre budgétaire constant, il nous faut plus que jamais mettre l’accent sur la qualité et l’efficacité de la dépense publique, aucun scrupule à mettre fin aux dépenses qui ne produisent pas les résultats attendus en matière d’insertion professionnelle. Je crois, à l’instar des sénateurs, à la force de l’évaluation des politiques publiques et des dépenses qui les sous tendent. L’efficacité de la dépense publique doit nous servir de principe directeur, même si nous devons évidemment prendre en compte l’effet récessif et l’effet emploi dans nos décisions de politique publique. Les baisses prévues en 2025 permettent de mettre à contribution de manière raisonnée raisonnée l’ensemble des structures qui contribuent au service public de l’emploi. Il est proposé, dans le budget qui vous est soumis, un équilibre entre nécessaire contribution au redressement des finances publiques et poursuite du soutien aux dispositifs qui marchent. En cohérence avec la feuille de route du Gouvernement en matière d’emploi et de travail, nous avons bâti ce budget autour de trois priorités. Il s’agit, premièrement, d’engager en faveur du retour à l’emploi des dépenses actives, tournées vers les dispositifs qui fonctionnent et qui ont prouvé leur efficacité.

L’arbre ne doit pas cacher la forêt : France Travail disposera bien des moyens nécessaires pour assurer les missions que lui assigne la loi du 18 décembre 2023. Il est ainsi proposé de maintenir stable, en 2025, la subvention pour charges de service public que l’État verse à France Travail, à hauteur de 1,35 milliard d’euros, conformément d’ailleurs aux engagements que l’État avait pris auprès de l’Unédic il y a quelques mois. Cet important de l’État est conforté par la hausse mécanique de la contribution de l’Unédic à France Travail en 2025. Ces moyens, qui sont également confortés par des efforts d’efficience et par des redéploiements, permettront de poursuivre la réforme pour le plein emploi. Le 1 janvier est à cet égard une étape importante. C’est la date à laquelle tous les nouveaux bénéficiaires du RSA, tous les flux entrants et tous les nouveaux jeunes accueillis en mission locale, seront inscrits comme demandeurs d’emploi, orientés, reçus et accompagnés de manière harmonisée, cohérente, mais aussi plus réactive et efficace, par l’opérateur le plus adapté. Mon ministère et

dans le cadre de l’IAE seront stabilisés à un niveau élevé entre 2024 et 2025, à hauteur de 1,5 milliard d’euros. Nous avons presque doublé le niveau de soutien public depuis 2018. Cet investissement public a permis de développer des structures nouvelles et d’augmenter de manière importante le temps de travail en insertion. Mais, après cette forte croissance, la stabilisation doit maintenant apporter de la lisibilité aux acteurs et accroître l’efficacité de nos interventions.

En premier lieu, et malgré un budget global en baisse, j’ai décidé de maintenir l’enveloppe prévue dans le projet de budget pour 2025 en faveur des pactes régionaux d’investissement dans les compétences, les fameux

En second lieu, je demande aux régions qui reçoivent ces fonds de renforcer encore davantage le fléchage de ces crédits vers les métiers en tension, vers les métiers nécessaires à notre souveraineté nationale et à la réindustrialisation de notre pays. Les services déconcentrés de l’État discuteront avec les exécutifs régionaux pour mettre à jour et recentrer la liste des métiers dont les formations sont financées par les Pric. Les formations au plus près des besoins des employeurs doivent être privilégiées ; encore une fois, le seul critère est celui de l’efficacité. Le soutien à l’emploi consiste également à accompagner les salariés et les entreprises lorsqu’elles sont en difficulté. À l’occasion de l’examen de ce projet de loi de finances, dans un contexte de hausse du nombre des restructurations

à se former pour être en mesure d’anticiper. Il s’agit véritablement d’adapter l’APLD aux réalités économiques du moment, sans rouvrir les vannes de la période du covid 19, mais en préparant mieux les transitions

prochaine. Mon deuxième axe est celui de la responsabilité budgétaire. Je suis convaincue de la nécessité du redressement de nos comptes publics, et ce d’autant plus que je suis responsable de la pérennité du financement de la protection sociale, que les salariés et les entreprises financent et sur laquelle ils comptent. Il ne s’agit pas de casser ce qui marche ! J’ai entendu certaines inquiétudes s’exprimer sur la question de l’apprentissage et du soutien afférent… Nous poursuivrons la révolution de l’apprentissage qui a été lancée en 2018. Nous changeons les modalités, les représentations

les besoins des entreprises. Nous avons lancé une concertation avec les partenaires sociaux et souhaitons remettre les branches au cœur du jeu afin qu’elles puissent mieux différencier la prise en charge des coûts de formation

dépassé, conformément à l’organisation de nos travaux décidée par la conférence des présidents et en accord avec la commission des finances, la suite de l’examen de cette mission serait reportée au samedi 7 décembre.

concernant le financement des formations à distance ou la prise en charge des dépenses de communication d’un certain nombre d’écoles. Telles sont les principales composantes de cette réduction supplémentaire. La

constitue un cadeau coûteux fait aux grandes entreprises, sans bénéfice clair pour les jeunes, dont l’entrée sur le marché du travail reste incertaine. Les experts sont unanimes quant à la nécessité d’une réforme. Dès 2023, l’économiste Bruno Coquet estimait qu’un meilleur ciblage des aides permettrait d’économiser jusqu’à 8 milliards d’euros.

Pantel. Le présent projet de loi de finances prévoit des ajustements du dispositif d’aide à l’embauche d’apprentis. Actuellement fixée à 6 000 euros par apprenti, cette aide constitue un levier essentiel pour encourager l’apprentissage, notamment dans nos petites entreprises. Or le Gouvernement envisage de réduire son montant à 4 500 euros,

Elles offrent aux jeunes leurs premières expériences professionnelles, souvent dans des métiers techniques ou manuels, indispensables à notre tissu économique. Réduire l’aide à l’apprentissage, c’est prendre le risque de fragiliser ces entreprises et de freiner l’accès des jeunes à l’emploi.

Par cet amendement, nous concentrons nos efforts sur les jeunes les plus exposés au risque de décrochage et sur les entreprises les plus engagées dans leur formation. L’amendement

persiste à ne pas répondre favorablement à cette revendication, et choisit de baisser le montant de l’aide en la maintenant pour toutes les entreprises. Du point de vue du Gouvernement, une entreprise du CAC 40 aurait donc, pour former un apprenti,

tout simplement pas l’apprentissage comme un vecteur de développement de nos entreprises et de promotion pour nos jeunes. Cette situation est particulièrement injuste pour les entreprises de proximité, qui forment les deux tiers des apprentis du pays

de la commission. Nous partageons l’idée de leurs auteurs : la diminution du niveau de la prime est une solution sous optimale par rapport à un meilleur ciblage des entreprises ou des apprentis éligibles. Nous ne sommes toutefois pas fermés, quant à nous, à une mesure intermédiaire négociée avec le Gouvernement, qui associerait une légère diminution du montant de la prime à un ciblage amélioré de l’aide.

devrait résulter un accroissement de 53 millions d’euros des recettes de France Compétences. Cet accroissement permet de minorer à due concurrence la dotation versée par l’État à l’opérateur.

avec les collègues d’Alsace Moselle et avec l’ensemble de la représentation nationale, parce que les efforts qui sont demandés le sont à toutes les entreprises de France. Pas

Nous avons beaucoup évoqué, durant l’examen de ce projet de loi de finances, la nécessité de rationaliser l’action publique, de la rendre plus efficiente. Il se trouve que le Gouvernement a proposé l’année dernière au Parlement de créer France Travail.

avis de la commission

que l’Apec travaille déjà en complémentarité avec France Travail et fait partie intégrante de ce nouveau réseau national pour l’emploi aux côtés des missions locales, de Cap emploi et d’un certain nombre

Mme la ministre.

pour animer une centaine de clubs, qui sont des relais précieux dans les entreprises privées pour la mise en œuvre de nos politiques de l’emploi. Ainsi, 1 500 événements sont organisés chaque année par ces clubs, par exemple des forums pour l’emploi, en lien avec les missions locales et avec France Travail.

Même si cette initiative a porté ses fruits dans certaines zones, les résultats de l’expérimentation demeurent contrastés à l’échelle nationale. Dans certains territoires, les effets positifs sont inexistants, en raison d’un manque de coordination et d’une faible adéquation entre les besoins locaux et les missions des entreprises à but d’emploi. En moyenne, le coût de l’accompagnement d’un salarié s’élève à plus de 20 000 euros par an, ce qui en fait l’un des dispositifs les plus

Cet amendement vise à revenir sur les conséquences de l’arrêté du 27 décembre 2023, qui a réduit de manière arbitraire la compensation due à l’Unédic au titre des exonérations de cotisations d’assurance chômage,

seraient, après montée en charge de la réforme, de 800 millions d’euros en 2026, puis de 400 millions par an. Ainsi les promoteurs du sérieux budgétaire, n’hésitant pas à déconsidérer les programmes économiques des autres forces politiques, sont ils également ceux qui, se servant allègrement dans les caisses de l’Unédic,

Le scrutin est ouvert.

par une baisse de 41,23 %, qui succède à une baisse de 24,5 % en 2024. Ainsi, ce sont 16 700 parcours emploi compétences (PEC) qui sont supprimés, déjà été en loi de finances pour 2024. La baisse du budget dédié aux contrats aidés absorbe 97,5 millions d’euros des 164 millions d’euros de coupes budgétaires en la matière Les besoins étaient déjà estimés à 612 millions d’euros l’an dernier, il faudra donc désormais 776 millions pour rétablir une véritable politique de l’emploi

cet amendement, nous proposons de rétablir une mesure essentielle pour faciliter le cumul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’une activité professionnelle. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoyait une enveloppe de 13 millions d’euros pour maintenir temporairement le bénéfice de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) aux allocataires de l’AAH 2 qui reprenaient une activité en milieu ordinaire, y compris au delà d’un mi temps. Ce dispositif devait permettre de sécuriser pendant deux ans le renouvellement des droits pour ces personnes, les encourageant ainsi à s’insérer ou à se maintenir dans l’emploi. Or cette disposition n’a malheureusement pas été mise en œuvre et a été annulée au printemps dernier. Cette suppression représente un recul pour l’accès à l’emploi des bénéficiaires de l’AAH qui souhaitent conjuguer activité professionnelle et protection sociale. Pourtant, ce type de mesure est essentiel pour lever les obstacles auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel. Il s’agit d’un levier d’autonomie et de participation active à la société, mais aussi de justice sociale.

sur les modalités d’articulation et de cumul entre AAH, revenus d’activité professionnelle et prime d’activité. Ce chantier ne pourra de toute façon pas aboutir à des mesures opérationnelles en 2025, chacun des minima sociaux

Or les mesures budgétaires prévues dans ce PLF pour 2025 sont largement en deçà de cette estimation. Je rappelle, notamment, votre volonté de supprimer 500 emplois à France Travail. Pis encore, les crédits destinés à des dispositifs fondamentaux, comme la formation des demandeurs d’emploi vulnérables ou les contrats aidés – nous venons d’en parler –, sont à la baisse dans le programme 102. Le service public de l’emploi a pourtant une mission essentielle : garantir un accompagnement effectif des des personnes les plus éloignées du marché du travail, dont les travailleurs en situation de handicap. Les retours du terrain montrent que, dans bien des cas, cet accompagnement est aujourd’hui insuffisant et manque d’efficacité.

Mme Monique Lubin. Cet amendement, auquel je tiens particulièrement, vise à mettre un terme à la dégradation du service public de l’emploi causée par l’externalisation de l’accompagnement et de l’insertion des personnes privées d’emploi.

De 250 millions d’euros de budget en 2018, celui ci est passé à 550 millions d’euros en 2022, puis à 650 millions d’euros en 2023. Avec France Travail, une nouvelle externalisation massive est prévue. Un accompagnement dédié à la reprise rapide d’emploi va être sous traité à des opérateurs privés. » Le recours à des prestataires privés représente un coût considérable pour l’opérateur du service public de l’emploi : près des deux tiers du budget dédié à la sous traitance, soit 1,6 milliard d’euros, sont allés aux prestations d’« accompagnement insertion » des personnes

voient leur chiffre d’affaires augmenter de plusieurs centaines de millions d’euros grâce à des financements publics. Ces montants proviennent en grande partie des cotisations des assurés sociaux, qui financent à 80 % le budget de France Travail la ponction sur l’Unédic décidée par l’État. Par exemple, une enquête de la CGT Chômeurs, relayée en juin 2024, révélait que la société Activ’Projet avait perçu 256 millions d’euros dans le cadre d’appels d’offres. Je pourrais continuer longtemps : de tels exemples sont légion. C’est particulièrement grave

de financements cumulés jusqu’en 2026, le présent projet de budget gèle les moyens de l’agence et entérine la suppression de 205 postes, après les modifications insuffisantes apportées en commission. Pourtant,

de cette mission va donc à contre courant des besoins de l’agence comme des enseignements de l’expérimentation ; il condamne ainsi les maigres effets positifs de la réforme du RSA, lesquels dépendent de l’accompagnement personnalisé et rapproché des bénéficiaires, ainsi que de la coordination des acteurs.

Les chiffres sont éloquents : alors que notre pays fait face à une croissance des défaillances d’entreprises et des plans sociaux, on envisage de réduire les moyens de notre service public de l’emploi.

Cette problématique est particulièrement criante dans les territoires ultramarins. À La Réunion, le taux de chômage atteint 16,8 %, contre une moyenne nationale de 7,3 %. Chez les jeunes, ce taux grimpe à 32 %. Dans ce contexte, réduire les effectifs de France Travail relèverait d’une décision incompréhensible. La diminution des effectifs, alors que le soutien à d’autres structures, comme les missions locales, est également en baisse, et alors que la réforme du RSA va engendrer un afflux d’inscriptions supplémentaires obligatoires à La Réunion, est inconcevable. Cet amendement vise donc à redéployer 25 millions d’euros de crédits pour préserver ces emplois, garantir un accompagnement de qualité et maintenir les ambitions de la loi pour le plein emploi. L’amendement

Dans ces conditions, les nouveaux objectifs pour 2025 semblent inatteignables, à moins d’une dégradation des actions qui risque de peser très négativement sur les personnes accompagnées. Pour toutes ces raisons,

la mission augmentent en réalité significativement par rapport à 2024 : la subvention pour charges de services publics budgétée sur le programme 102 est orientée à la hausse – 1,35 milliard d’euros, soit 100 millions d’euros de plus par rapport à 2024 de même que les transferts en provenance des programmes 102 et 103, qui s’établissent à 2,65 milliards d’euros pour 2025. Les crédits alloués par l’État à France Travail connaîtraient donc une hausse de 15,2 % entre la loi de finances initiale pour 2024 et le présent projet de loi.

Madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme du temps imparti pour l’examen de la mission « Travail, emploi et administration des ministères sociaux ». Il nous reste soixante et un amendements à examiner. conformément à l’organisation de nos travaux décidée par la conférence des présidents et en accord avec la commission des finances, la suite de l’examen de cette mission est reportée au samedi 7 décembre, à l’issue de l’examen des missions de la journée. Mes chers collègues,